d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce quinquennat, qui devait révolutionner la politique, s'abîme, semaine après semaine, dans des débats hystérisés pour faire oublier le fondement des injustices : des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. pauvres. En dix ans, le patrimoine des milliardaires a augmenté de 439 % dans notre pays. À ce rythme, le SMIC serait à 4 805 euros par mois

Vous répondez depuis des mois par une pirouette démagogique qui masque mal des objectifs violemment antisociaux. Depuis des décennies, le thème de la sécurité et la menace de l'immigration sont agités en permanence pour écarter la population du vrai débat qui décide de son destin collectif ? Avec quels moyens ? Monsieur le Premier ministre, après la loi sur le séparatisme et la loi pour une sécurité globale, qui confond le respect du droit à vivre en sécurité et la remise en cause systématique des libertés publiques, nous découvrons chaque jour de nouveaux projets de loi, en réaction à tel ou tel drame. Ce dont vous ne parlez pas, c'est la mise en cause des chômeurs, c'est la menace persistante de la réforme des retraites, c'est la casse continue du droit du travail. Monsieur le Premier ministre, la France est inquiète, non pas de l'autre, du voisin, de ceux qui viennent mourir sur les plages d'Europe, mais de l'avenir incertain de ses enfants et de cette profonde insécurité sociale, car le libéralisme détruit la solidarité et l'égalité. La crise a montré une chose : notre pays et l'Europe sont riches et peuvent disposer de moyens considérables pour agir. Les centaines de milliards d'euros dont vous disposez pour faire face à cette crise, fruit de l'activité humaine, serviront-ils au ou, pis, à achever notre modèle social ? Ou bien serviront-ils à rebâtir une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement ?

le grand pays de la zone euro qui a perdu le moins d'activité depuis le début de la crise, d'après les chiffres d'Eurostat et de la Banque de France. Nous avons collectivement résisté. On peut dire que ce n'est pas assez

et le redémarrage de notre pays et de notre économie. Tout le Gouvernement est mobilisé à cette tâche.

I-ni-ma-gi-nable ! Pourtant, il l'a fait ! Non, je ne parle pas ici d'un exploit sportif ou d'un geste héroïque hors norme. Il y a malheureusement longtemps que l'audace n'est plus l'apanage des seuls héros. héros. Je parle ici de l'incroyable acte de piraterie aérienne d'État ordonné dimanche dernier par M. Loukachenko, l'inaltérable président-autocrate du Bélarus. En apprenant la nouvelle, j'ai un instant cru à un canular. Aujourd'hui encore, je me demande quel degré de folie peut expliquer une telle violation du droit international, dans l'unique but de procéder à l'arrestation d'un jeune journaliste. Je ne suis visiblement pas le seul à avoir été sidéré, si j'en juge, monsieur le ministre, par la fermeté de votre réaction dès dimanche après-midi. Avant-hier, des sanctions européennes inédites ont été prises face à cet acte d'une gravité encore plus inédite. Comme le reconnaissait hier le Président Macron à l'issue du Conseil européen, « la politique des sanctions progressives sur des situations gelées n'est plus une politique efficace ». Il s'interrogeait sur les limites actuelles des sanctions, sans tomber dans l'engrenage d'un possible conflit armé. armé. Ma question, monsieur le ministre, est donc simple : sommes-nous vraiment au bout des sanctions applicables au Bélarus ? Ne peut-on élargir les sanctions à quelques centaines, voire quelques milliers d'autres responsables biélorusses ? ? Nous le savons, ce régime ne repose plus que sur quelque 10 000 cadres qui en tirent directement profit. Par ailleurs, il faut absolument veiller à ce que cet acte de piraterie pas la voie à des actes similaires dans d'autres espaces aériens sensibles. Aussi, je voudrais savoir si la France est prête à demander l'activation de l'article 88 de la Convention de Chicago, afin de suspendre les droits du Bélarus au sein de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La parole

dans leur comportement déstabilisateur et répressif. Vous l'avez souligné avec raison, le Conseil européen de lundi soir a réagi avec une très grande fermeté et une très grande unité. Les mesures prises lundi soir sont applicables dès aujourd'hui. Je pense en particulier aux dispositions relatives au domaine aérien, avec l'interdiction d'utiliser l'espace aérien européen et de se poser dans les aéroports européens pour toutes les compagnies du Bélarus. Je pense aussi à l'interdiction, pour les compagnies européennes, de survoler le Bélarus. Vous me demandez si l'on va aller plus loin. La réponse est « oui ». prises par le Conseil lundi soir, il a été demandé à la Commission de préparer une panoplie de sanctions supplémentaires par rapport aux 88 sanctions déjà prises au moment des élections truquées d'août dernier. Je me suis entretenu

donc de leur bon déroulement démocratique et de leur impartialité. Pensez-vous que votre annonce de poursuites pénales contre une candidate à une élection qui avait simplement émis une opinion sur votre action soit compatible avec vos fonctions ? Confirmez-vous cette annonce

je vous ai écouté avec attention. Sur le fond, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, nous devons protéger avec force les policiers qui nous protègent : nous le pensons, nous le pensons, nous le disons, et nous l'avons fait quand nous étions au pouvoir. Je vous ai demandé solennellement de nous dire ce qui vous a autorisé à tenter d'intimider une candidate, vous qui, au contraire, avez la charge de protéger la parole libre et démocratique de Mme Pulvar, comme de toutes celles et de tous ceux qui concourent aux élections. Pourquoi avoir créé une polémique de plus, alors que votre rôle est de garantir le débat apaisé dont notre démocratie a, plus que jamais, besoin ? Pourquoi, dans ce moment de montée de toutes les violences et tensions, préférez-vous créer de l'agitation et du désordre, par des opérations de communication et de saturation médiatique, alors que les citoyens attendent de vous une action efficace, de la stabilité et de la cohésion ? Ce que nous demandons, nous, parlementaires, c'est que vous commenciez, vous, par respecter notre État de droit et la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ainsi que la sérénité que votre fonction exige pour protéger nos concitoyens.

monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, dans un tout autre registre. Comme chaque année dans le Var à l'approche de la saison estivale, la même question revient : y aura-t-il un Dragon 83 affecté à notre département cette année ? S'il s'agit de détacher un hélicoptère de la sécurité civile sur la base du Luc-en-Provence, il semblerait que, cette année, outre le manque global d'appareils de ce type, se pose le problème de leur maintenance et de la disponibilité de leur équipage. D'où l'angoisse des Varoises et des Varois, mais aussi celle des habitants du département de la Gironde, qui voient leur Dragon 33 surchargé par le non-déploiement d'un hélicoptère de la gendarmerie. Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre : quelles décisions comptez-vous prendre pour mieux préparer la saison 2021 en termes de moyens aériens en général ? le « en général », car ma question cache un besoin bien plus vaste lié à l'insuffisance du nombre d'appareils volants destinés à la lutte contre les incendies de forêt. Je veux parler du manque d'avions bombardiers d'eau amphibie, les fameux Canadair, capables d'écoper en mer ou sur toute autre étendue d'eau.

Chaque année, confrontées à des chaleurs caniculaires, les forêts du sud de la France, mais aussi celles du Portugal, de l'Espagne et, tout récemment, de la Grèce - et j'en oublie -flambent, ce qui occasionne des dégâts irréversibles sur l'environnement, la biodiversité et le dérèglement climatique. Aussi, cadre de la prochaine proposition de loi sur la sécurité civile, dite « Matras », et du plan de relance, ne pourrait-on pas envisager une véritable stratégie d'acquisition ou de fabrication de ce type d'appareil à l'échelle européenne ?

de redire à quel point nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et tous ceux qui concourent à la sécurité civile de notre pays sont indispensables. Leur courage mérite d'être soutenu, et je sais que vous le faites.

à la lecture de ses orientations. Malgré un débat public sur la PAC montrant clairement les attentes en matière de transition agricole et alimentaire, malgré les alertes d'organisations agricoles et environnementales, dont la plateforme Pour une autre PAC, relayées par des parlementaires, malgré l'ensemble des signaux pointant l'urgence écologique, le ministre a choisi d'opter pour une PAC du quasi-, qui du quasi-, qui fige à la fois les inégalités existantes et un modèle dont on sait aujourd'hui pertinemment qu'il n'est ni durable, ni créateur d'emploi, ni rémunérateur, ni conforme aux attentes des citoyens.

chargé de conseiller le Premier ministre avait fait de la PAC, dans son rapport, un levier de la transition agroécologique. Il avait également estimé que l'agriculture biologique était la plus performante en termes tant économiques qu'environnementaux. Après avoir supprimé le financement national de l'aide au maintien,

d'abord de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Julien Denormandie, qui est actuellement à Bruxelles pour le Conseil européen. Il aurait aimé tordre le cou à une rumeur qui circule depuis quelques jours : non, le soutien à l'agriculture biologique ne diminue pas ! Au contraire, les aides augmentent, et fortement. Nous

Oui, monsieur le sénateur, nous assumons totalement le fait de vouloir faire du bio une filière agricole française d'excellence, avec toujours plus d'agriculteurs qui s'y consacrent. Ne voyons pas les choses en petit, en nous focalisant sur les seules aides au maintien. Ayons au contraire une logique conquérante pour le bio, en favorisant les aides à la conversion. N'ayons pas peur d'être ambitieux pour les 400 000 agriculteurs français, n'ayons pas peur d'accompagner, d'inciter et de convaincre des bienfaits de l'agroécologie. Tel est le sens de l'investissement de 1,2 milliard d'euros pour la transition agricole dans le plan de relance. Notre conviction est intacte : nous préférons « embarquer » plutôt qu'imposer ; nous préférons réussir plutôt que brimer. Nous construisons la transition agricole avec les agriculteurs, nous menons de front la bataille du bio avec eux et avec des moyens hier dans les pages d'un quotidien, nous forgeons une agriculture respectueuse des hommes, des animaux et de la terre. Nous le faisons avec les agriculteurs, et pas contre eux.

monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Vous le savez, une attaque informatique a paralysé un oléoduc majeur de la côte est des États-Unis. Les infrastructures d'énergie sont des cibles privilégiées des cyberattaques, au regard des graves effets que cause leur mise à l'arrêt. Afin de moderniser ces infrastructures, le président Biden a annoncé un plan de 2 000 milliards de dollars, dont 20 milliards seront dédiés à la cybermodernisation des réseaux électriques. Un nouveau crédit d'impôt financera les cybertechnologies de ces réseaux. La France n'est malheureusement pas à l'abri de ces menaces, qui prolifèrent tous azimuts. Après les scandales Cambridge Analytica visant à influencer le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump, notre pays a été le théâtre de manoeuvres de déstabilisation lors des dernières élections présidentielles. Ces actions perturbent notre vie démocratique, ainsi que notre vie sociale et économique. Des hôpitaux ainsi que des médias français ont subi des cyberattaques. Plusieurs en ont été réduits à revenir au mode papier et stylo. Dans le même objectif de déstabilisation, certains influenceurs ont récemment été approchés, afin de participer à une campagne de désinformation sur le vaccin Pfizer. Les commanditaires, probablement russes, cherchent à perturber la vaccination et, donc, la reprise de l'activité dans notre pays, en instillant une défiance à l'égard des scientifiques.

Néanmoins, restons lucides : le nombre de cyberattaques visant notre pays a été multiplié par quatre entre 2019 et 2020. Dans un contexte international troublé, notamment aux frontières de l'Union européenne, et à l'approche des élections de 2022, la France est-elle prête, madame la secrétaire d'État, à faire face à l'intensification de ces attaques ? Quelles mesures sont prises, notamment en matière de recherche et de formation, pour renforcer la résilience de notre pays face aux cyberattaques ? La parole

des cybermenaces. Aujourd'hui, le cyberespace est un espace de conflictualité de plus en plus important, dans lequel les menaces augmentent chaque jour. Entre 2019 et 2020, selon l'Anssi, le nombre de victimes de cyberattaques a été multiplié par par quatre. Je crois que ce chiffre parle de lui-même. Si la sécurisation des systèmes d'information doit être évidemment une priorité, toutes les organisations doivent aussi intégrer la possibilité de subir une cyberattaque et, donc, se mettre en capacité d'y répondre. C'est la définition même de la résilience dans le cyberespace. Cette nécessité est totalement identifiée dans le cadre de la stratégie d'accélération Cyber qui a été annoncée le 18 février dernier par le Président de la République et est financée à hauteur de 1,4 milliard d'euros.

et innovantes de cybersécurité ; le renforcement des liens et des synergies entre les acteurs de la filière ; le soutien à la demande ; le renforcement de l'offre de formation des jeunes et des professionnels à ces métiers émergents de la cybersécurité ; le soutien en fonds propres au développement des entreprises de la filière un effort spécifique en faveur de la cybersécurisation des établissements de santé. Plusieurs actions concrètes, madame la sénatrice, ont déjà été mises en oeuvre. Premièrement, sans attendre cette augmentation des cyberattaques, nous avons en permanence, depuis 2017, augmenté les moyens humains de l'Anssi. Un appel à manifestation d'intérêt a par ailleurs été lancé en direction des collectivités, des établissements de santé et des ports afin de mettre en place des démonstrateurs de cybersécurité adaptés aux besoins de ces structures spécifiques. L'Anssi a commencé à mettre en oeuvre un plan de sécurisation des administrations

Votre question se pose- le Gouvernement en est conscient -, le plan se déroule et nous sommes très attentifs à ce sujet des cyberattaques. La parole

un enfant de 5 ans, grièvement blessé alors qu'il traversait à vélo sur un passage protégé ; plus récemment, à Lyon, une femme fauchée par deux jeunes à scooter pas une semaine ne passe sans que les agissements, aux conséquences parfois tragiques, des auteurs de rodéos motorisés fassent la une des médias. Les victimes se multiplient. Les nuisances, pour les riverains, s'accumulent et instaurent un climat de violence. Malgré la loi du 3 août 2018, qui fait de cette pratique un délit puni d'une peine d'emprisonnement allant de un à cinq ans, le phénomène perdure et s'amplifie. En cause, l'application de ce texte, qui se heurte à plusieurs limites. Tout d'abord, concernant les directives données aux policiers, la consigne est de ne pas aller au contact des contrevenants par peur de provoquer des accidents ou des émeutes urbaines. L'affichage de fermeté du Gouvernement bute ici sur la réalité des faits. Si l'on comprend bien les difficultés inhérentes à ce type d'interventions, une telle consigne n'en demeure pas moins un redoutable aveu d'impuissance. Conséquence majeure et regrettable : le sentiment que certains individus ne sont pas tenus de respecter les lois de la République. qui est du type de sanctions appliqué, la confiscation des véhicules est aujourd'hui la mesure la plus efficace pour lutter contre cette pratique dangereuse ; pourtant, sa mise en oeuvre n'est pas systématique et semble même marginale. Cela pose de sérieuses questions quant à la capacité des autorités à lutter contre les récidives, en particulier lorsque les engins saisis sont ensuite restitués aux fauteurs de troubles. Enfin, récemment, l'État a été condamné pour son inaction à faire cesser ces rodéos motorisés, preuve, s'il en était besoin, que la loi n'est pas exécutée comme il le faudrait. L'ensemble de ces observations, liées tant à la persistance de ces pratiques qu'à la faiblesse de l'État là où il s'agit de faire respecter la loi, crée un sentiment de totale impunité qui est incompatible avec la légitime attente de sécurité qui émane de nos concitoyens. Monsieur le ministre, face à ce constat d'échec, quelles actions envisagez-vous de mener pour lutter contre ce fléau ? La parole

les événements incriminés ; elle ne couvre pas des faits qui nous seraient imputables. Voilà pour la précision ; elle est toujours utile. Par ailleurs, depuis la promulgation

accordé à la justice, permet la mise en oeuvre de saisies immédiates de scooters. Je vous indique d'ailleurs que j'ai demandé à l'ensemble des maires de notre pays

J'ajoute que j'ai pris une circulaire reprenant les 350 infractions dites « de basse intensité »- j'exclus bien sûr les homicides involontaires, dont vous avez parlé

de l'emploi et de l'insertion, dans un rapport publié mardi dernier, la Cour des comptes certifie les comptes 2020 de plusieurs branches du régime général de la sécurité sociale moyennant « un nombre accru de réserves ». Et c'est tout particulièrement la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui est la cible de critiques, du fait d'erreurs toujours plus nombreuses dans le calcul des prestations de retraite. Une prestation sur six nouvellement attribuée ou révisée en 2020 a comporté au moins une erreur financière, et ce, dans la grande majorité des cas, au détriment des retraités Concrètement, l'impact cumulé dans le temps de ces erreurs est estimé à 1,6 milliard d'euros et, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse elle-même, la moitié des retraités lésés ont subi un préjudice égal ou supérieur à 123 euros par an. Ces sommes sont loin d'être négligeables, surtout quand on sait que la pension moyenne versée aux retraités en 2019 était de 1 393 euros net mensuels. Certes, madame la ministre, ces erreurs ne sont pas nouvelles, mais la situation se dégrade année après année. D'une erreur sur neuf dossiers il y a cinq ans, nous en sommes dorénavant à une erreur sur six dossiers Il y a deux mois, des retraités manifestaient pour une revalorisation de leur pension. On comprend donc que la révélation de ces erreurs de la caisse de retraite soit mal vécue, d'autant que celles-ci concernent prioritairement les personnes les plus modestes. La Cour des comptes relève que ce sont en effet les pensions les plus faibles qui sont touchées, le taux d'erreur étant de près de 23 % pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Madame la ministre, ma question est extrêmement simple : comment redonner confiance à nos concitoyens et améliorer la fiabilité du système ?

une réalité. Elles ont augmenté ces dernières années- vous l'avez dit : en 2020, elles concernent une pension sur six, contre une pension sur neuf en 2016. Cela n'est pas négligeable. L'erreur médiane est en défaveur des assurés : elle est de l'ordre de 10 euros par mois. Je rappelle tout d'abord que le calcul des pensions est un exercice extrêmement complexe, d'autant qu'il existe 42 régimes dépendant des statuts personnels. Pour calculer une pension de retraite à l'euro près, il ne faut oublier aucun élément de la vie professionnelle et intégrer les données et règles d'interaction avec les autres régimes de retraite. Avec la complexification des carrières, cette mission devient de plus en plus exigeante. L'assurance retraite fait déjà un travail considérable pour que ces erreurs soient détectées et corrigées. C'est d'ailleurs l'une de ses activités principales. Grâce à ce travail, au moins 40 % des anomalies sont corrigées dans les semaines et mois qui suivent leur identification, selon l'assurance retraite. Il est donc essentiel que ce travail du quotidien soit encore renforcé et que ces anomalies soient traitées plus en amont. C'est pourquoi l'assurance retraite a mis en place un plan d'action global qui doit permettre à court terme, mais aussi à moyen et long termes, de mieux comprendre les sources des anomalies pour les identifier et y apporter des traitements adaptés, de renforcer la supervision et la formation internes, de développer de nouveaux outils informatiques. Les services de l'assurance retraite sont pleinement mobilisés, soyez-en assurés. Élisabeth Borne et Laurent Pietraszewski sont très attentifs à ce que ce plan ait des effets concrets dès cette année. La parole

Il n'y a pas si longtemps, nous vivions la crise des gilets jaunes. Ces manifestations ont révélé les tensions et les fractures à la fois sociales, économiques et territoriales qui minent notre société. de covid et les confinements successifs ont mis un frein à l'ensemble des mouvements sociaux en faisant rentrer à la maison toutes les contestations. Cependant, les reproches à l'égard de votre politique sont toujours présents et se sont amplifiés. Alors que nous sortons progressivement de la crise sanitaire, il faut regarder les choses en face : depuis que votre gouvernement est en place, le quotidien des classes populaires ne s'est pas amélioré. Dans nos territoires, on constate chaque jour un éloignement grandissant et très inquiétant entre les Français ruraux modestes et la politique menée. Vous leur demandez de prendre le vélo et les transports en commun, de bazarder le diesel pour l'électrique, d'abandonner les chaudières au fioul. Quoiqu'elles soient dictées par de bonnes intentions, ces mesures sont éloignées des préoccupations et du quotidien de nombreux Français. Attention au choc en retour, car vous les sommez de s'adapter ! Malgré le « quoi qu'il en coûte », qui draine en masse l'argent public, la France populaire n'y trouve pas son compte. Nos concitoyens les plus modestes ont toujours l'impression de travailler durement sans gagner leur vie dignement. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience de cette France-là, qui gronde, peine et ronge son frein ? Avez-vous conscience que la plus petite décision malvenue, prise au mauvais moment, peut raviver la violente contestation que ni vous ni nous ne souhaitons ? En conclusion, ma question est simple : que comptez-vous faire pour réduire cette fracture sociale et territoriale si évidente

nous avons fait tenir. Le Gouvernement n'a pas fait que soutenir l'économie- je pense aux différentes aides exceptionnelles et légitimes qui ont été déployées en faveur des plus fragiles et qui sont déjà mises en oeuvre.

Au-delà de leur ampleur, il est important de dire que ces aides atteignent leur cible. Une étude du Trésor, fin 2020, démontre clairement que les deux tiers des bénéficiaires des aides débloquées pour les ménages sont parmi les 20 % des Français les moins riches. J'ajoute

les catégories populaires, nos concitoyens les plus fragiles, sont au coeur de nos préoccupations depuis le début de ce quinquennat en 2017. Ah bon ! Nous n'avons pas attendu la crise

que nous travaillons à l'augmentation du pouvoir d'achat des plus fragiles et nous avons bien l'intention de continuer. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la question des déserts médicaux est toujours d'actualité dans notre pays. Des millions de personnes éprouvent des difficultés à consulter un médecin généraliste ou un professionnel de santé de premier recours. de premier recours. Beaucoup de collectivités territoriales ont pris et prennent des initiatives en ce domaine afin de résoudre cette injustice territoriale. Ici, au Sénat, voilà deux ans,

la disposition qui avait été proposée à l'époque par la sénatrice Corinne Imbert. La question du défi démographique et de la désertification médicale ne date pas de cette semaine- vous l'avez rappelé ; elle ne date pas non plus de ce quinquennat

généralistes et spécialistes en accès direct a effectivement baissé depuis de nombreuses années. Ce gouvernement en a fait l'une de ses priorités : un certain nombre de mesures ont été adoptées depuis le début de ce quinquennat- je ne vais pas toutes les énumérer ici. Ce n'est pas la question ! Je

dans la lignée du dispositif que vous évoquez : la création de 4 000 postes d'assistants médicaux pour seconder et appuyer les médecins dans leurs tâches administratives et soignantes, le déploiement de 600 médecins généralistes dans des territoires prioritaires, dont 200 priorisés sur les territoires ruraux, en exercice partagé

le secrétaire d'État, merci pour toutes ces considérations ; peut-être mes oreilles entendent-elles mal, mais je n'ai pas entendu quand ce décret serait publié. Et je trouve tout de même problématique

Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, Stéphanie, jeune maman, est abattue lâchement en pleine rue par son compagnon, réfugié, fraîchement sorti de prison. Dans l'Essonne, une femme est tuée de plusieurs coups de marteau à la tête devant son fils de 11 ans.

je sais combien le sujet des violences conjugales est un sujet qui vous est cher, sur lequel vous vous êtes longtemps investie. Je vous remercie de votre question : longtemps, trop longtemps, notre société a été sourde aux cris d'alarme, aveugle aux souffrances et muette face aux violences qui étaient faites aux femmes et aux filles. Comme vous le savez, le Gouvernement et la majorité se sont mobilisés depuis 2017 pour enrayer ce fléau. Cette mobilisation générale s'est traduite par le vote de quatre lois en quatre ans et de quarante-six mesures issues du Grenelle des violences conjugales, parmi lesquelles les ordonnances de protection, qui ont été démultipliées,

de pouvoir répondre à toutes les femmes qui sont victimes de violences dans notre pays, qu'elles se trouvent dans les territoires ultramarins ou dans l'Hexagone, qu'elles soient ou non malentendantes, sourdes ou aphasiques.

Nous demandons l'augmentation du budget des bracelets ? Vous vous y opposez. Nous demandons de la fermeté ? Vous libérez des conjoints violents faute de places de prison- 15 000 places promises, 1 500 seulement aujourd'hui construites. La non-exécution des peines se fait au détriment des Françaises et des Français. Vous voulez redorer la « grande cause du quinquennat » qu'est l'égalité entre les hommes et les femmes est-ce redorer cette grande cause que de s'opposer aux mesures innovantes et adaptées aux réalités actuelles que nous proposons ? Nous avons demandé que les réfugiés soient déchus de leur statut lorsqu'ils commettent des crimes et délits, notamment des violences conjugales ? Rejeté

Est-ce au nom des valeurs du sport et de la République que votre collègue ministre des sports ne s'oppose pas, loin de là, à ce que des signes qui constituent un interdit de liberté, d'égalité et de fraternité, comme le hijab de sport, soient promus ? Il y a quelques jours, cette même ministre ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'un chanteur représente l'équipe de France de football tout en chantant notamment l'agression sexuelle de personnalités politiques ! Où est la cohérence au sein de votre gouvernement ? Beaucoup de paroles, beaucoup de communication ; mais la grande cause du quinquennat, ... Il faut conclure. ... loin d'être redorée, se perd dans les méandres du « en même temps » et parfois même du séparatisme. C'est vraiment regrettable

mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis dix-huit mois, la commission des lois et la commission des affaires sociales du Sénat travaillent sur les questions d'irresponsabilité pénale et d'expertise psychiatrique. et d'expertise psychiatrique. Nous avons, hier, adopté un texte. Les réflexions du Gouvernement, celles de l'Assemblée nationale, sur cette question de l'irresponsabilité sont des réflexions pour l'avenir. Je voudrais, moi, vous parler de la situation présente.

de quelles mesures de soin ou d'accompagnement bénéficient les personnes concernées ni, d'ailleurs, s'ils en bénéficient, qui ils sont et où ils demeurent. Comment entendez-vous assurer le suivi des auteurs irresponsables alors que vous avez supprimé la collecte de ces données ? Par dépêche du 18 juin 2019, la direction des affaires criminelles et des grâces a informé les juridictions de sa décision de supprimer le dispositif de recensement des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par souci d'alléger leur travail. La dernière étude épidémiologique générale réalisée en France sur la santé mentale dans les prisons remonte quant à elle à 2007 ... Monsieur le Premier ministre, voilà ma question : où en êtes-vous de la mise en place du système de remplacement de la collecte et du suivi des personnes irresponsables ? comptez-vous, sans ces données, assurer la sécurité des Français ?

Mais vous ne souhaitez pas le circonscrire à la discussion que nous avions : vous voulez savoir quel est le sort qui est réservé à ceux qui sont déclarés irresponsables. Nous avons effleuré cette question hier vous devriez poser la question au ministre de la santé, pardonnez-moi de vous le dire, car, à compter du moment où un homme est déclaré irresponsable, il n'est pas détenu : il est soigné.

Pour le reste, la décision du 14 avril nous a beaucoup émus. Certains de nos compatriotes n'ont pas compris cette décision. Elle a été rendue en droit, et les juges ont pris soin de préciser qu'ils ne pouvaient pas distinguer là où la loi ne le permettait pas. Vous avez tenté de remédier à cela ; j'ai moi-même, à la demande du Président de la République, travaillé à un texte. J'ai reçu les cultes, les magistrats, des avocats, des psychiatres, et j'ai souhaité

il inverse les termes de la politique de l'offre et de la demande et positionne les acteurs du service public de la culture dans une concurrence directe et frontale avec les grands opérateurs du privé et avec les industries culturelles du loisir. Le projet de pass culture part d'un principe jamais débattu en vertu duquel la question de l'accès à la culture des jeunes est d'abord un problème économique et technologique avant d'être un sujet éminemment symbolique et politique, dont l'exclusion sociale et territoriale est le marqueur principal. Le projet de pass culture ignore l'engagement quotidien des équipes de médiation et de transmission culturelles, dont je rappelle qu'il est financé très majoritairement par les collectivités territoriales. Le projet de pass culture draine sur lui un budget intarissable, « quoi qu'il en coûte », véritable gabegie dont il ne fait nul doute que la Cour des comptes en dénoncera les errements le moment venu. Après Françoise Nyssen et Franck Riester, Roselyne Bachelot est la troisième ministre à récupérer ce mistigri présidentiel. À l'heure où la généralisation du pass culture vient d'être décidée par le Président de la République lui-même, sont-ce McFly et Carlito qui en assureront le service après-vente, ou ne pensez-vous pas plutôt qu'il est grand temps d'arrêter les frais ?

du déploiement et de la généralisation du pass culture, porté par le Président de la République et par ma collègue Roselyne Bachelot dès vendredi dernier, montrent que plus de 650 000 jeunes ont téléchargé l'application : c'est

elle ne convainc pas grand monde ici. En tout point du pays, c'est la puissance du réseau de la culture décentralisée qui assure la relation au public jeune, en particulier. C'est une action durable constante, dont les artistes sont les premiers acteurs. La priorité à accorder à la jeunesse ne saurait passer par des gadgets décidés verticalement depuis Paris, au mépris des réalités de nos territoires.

Il y a deux ans est né en Algérie un mouvement citoyen, pacifique et mixte, qui constitue un immense espoir pour la jeunesse algérienne. Ce mouvement, que demande-t-il ? Un pouvoir civil, des libertés démocratiques, un meilleur partage des richesses et la fin de la corruption. Bref, un avenir. Depuis quelques mois, à la faveur de la crise sanitaire, la répression s'est abattue sur ce mouvement. On ne compte plus les citoyens, les militants, les journalistes arrêtés, emprisonnés, condamnés.

Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire pour les garantir en Algérie ?

et elle s'exprime au plus haut niveau, puisque le président Abdelmadjid Tebboune et le président Macron se parlent régulièrement. Le Premier ministre se rendra bientôt à Alger pour un comité interministériel de haut niveau, qui devait avoir lieu il y a quelques jours, mais qui a été repoussé en raison de la pandémie.

et avec dignité, lors du Hirak. Notre seul souhait, c'est la réussite des réformes au bénéfice de l'Algérie et des Algériens. En effet, madame la sénatrice, c'est aux Algériens, et à eux seuls,

ce pays pour délit d'opinion. Le processus que vous décrivez, celui de la réforme en profondeur de l'Algérie par la démocratie, est un processus idéal. C'est celui dont nous rêvons tous, mais il n'a pas lieu ! Ce qui se passe actuellement en Algérie est l'inverse d'un processus de réforme. Vous savez bien que les atteintes quotidiennes aux libertés sont extrêmement sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de ce pays. La jeunesse algérienne est aujourd'hui sans avenir ; elle le sait, elle le ressent. Aussi, que se passe-t-il ?

Ce qui se passe en Algérie, c'est notre coeur qui le ressent

Madame la secrétaire d'État, le 8 avril dernier, les langues régionales ont obtenu une reconnaissance et une victoire historiques à l'Assemblée nationale. La loi proposée par notre collègue député Paul Molac a en effet été adoptée à une très large majorité, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, avec 276 voix pour et seulement 76 voix contre. Ce vote est le résultat d'un processus démocratique et transpartisan pour la promotion des langues régionales, notamment grâce à l'article 4, qui inscrit dans la loi l'enseignement immersif. Pourtant, le Gouvernement a décidé de s'y opposer en déposant un recours devant le Conseil constitutionnel, contre sa propre majorité. Et- faut-il y voir un message symbolique ? -, c'est le 21 mai, date de la Journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et et signé ce qui ressemble à l'arrêt de mort des langues de France, en censurant l'essentiel de la loi Molac dans des conditions on ne peut plus troubles. En effet, plusieurs députés La République En Marche ont publiquement affirmé que leur signature sur ce recours leur avait été arrachée et ont écrit au Conseil constitutionnel pour la retirer. En même temps, le Premier ministre, hier, et le Président de la République, aujourd'hui, déclarent que « les langues régionales sont une chance pour la République ». Pour minimiser l'effet de cette censure, on annonce la création d'une énième mission, confiée à deux députés. Qu'attendez-vous concrètement de cette mission ? Ma question est simple : quel est l'avenir des écoles publiques et associatives basques, bretonnes, alsaciennes, occitanes et autres, sous contrat avec l'État ?

En toute hypothèse, je rappelle au Sénat que la principale censure prononcée par le Conseil constitutionnel l'a été

Vous êtes, madame la sénatrice, une élue de l'Alsace. Je suis moi-même élu d'une région où les langues régionales sont très développées. Renseignez-vous : je les ai toujours soutenues et encouragées.

de cette décision et d'en tirer tous les enseignements. Nous le ferons avec la volonté de préserver et de maintenir le rôle des langues régionales à l'école, dans le cadre de l'unité de la République.

Après que les deux députés m'auront rendu leurs conclusions, je l'ai dit, je recevrai l'ensemble des associations concernées, pour que, sereinement, pour que, sereinement, nous en tirions toutes les conséquences. Ces dernières, je l'indique également au Sénat, seront marquées par la volonté politique du Gouvernement de préserver la richesse que constituent, dans le cadre de l'unité de la République, les langues régionales.

filiale française du plus gros américain. Contre une imprimante gratuite et 6 euros par mois et par pharmacie, toutes les données médicales de nos concitoyens sont automatiquement transmises : numéro de sécurité sociale, prénom, âge, sexe, affections, traitements, etc. Un « plat de lentilles » à l'échelle des profits suscités par ces données, qui sont ensuite revendues à toutes sortes de sociétés, qui, les États-Unis, peuvent ainsi faire du ciblage publicitaire de plus en plus précis, en justifiant un pseudo-intérêt d'ordre public qui ne peut être contrôlé. À ce jour, la moitié des pharmacies pratiqueraient cette collecte, soit 10 000 officines, et 40 millions de Français seraient ainsi concernés. Et cela en toute illégalité, puisque le règlement général sur la protection des données, le RGPD, impose une information préalable et l'expression d'un accord explicite explicite avant toute collecte de données. Or, en pratique, l'information n'est jamais affichée, et le consentement jamais donné. Plus grave encore, cette pratique serait connue du Président de la République et couverte au plus haut de l'État. Monsieur le secrétaire d'État, que pouvez-vous nous dire de ces méthodes ? Confirmez-vous qu'elles sont illégales ? Et si oui, qu'allez-vous faire pour mettre fin à la marchandisation de la santé des Français, qui ignorent cette pratique ?

que vous avez relayées et auxquelles il est important d'apporter des réponses précises, tant ces sujets sont importants pour nos concitoyens et pour nos libertés. Cette question porte sur l'accès aux données de santé de nos concitoyens par les pharmaciens et sur l'usage qui en serait fait, notamment par Iqvia.

Ces données permettent de mener des études d'intérêt public, qui visent, par exemple, à l'évaluation de la bonne utilisation du médicament, l'analyse scientifique et statistique des phénomènes liés à la persistance, la conformité, le respect des prescriptions et des contre-indications. Je précise que vous pouvez consulter ces études en ligne de façon transparente.

contrairement à ce que vous laissiez entendre, à la déclaration faite à la CNIL, laquelle prévoit que ces données traitées en interne ne sont pas transmises à des tiers. La CNIL avait souligné, dans son arrêt de 2018, l'intérêt public majeur que représentaient les études menées sur la base

Le dossier pharmaceutique, dont le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est responsable, et le dossier médical partagé sont totalement indépendants, là aussi, de la relation entre le pharmacien et la société. Il n'y a aucun accès possible de cette société à la carte Vitale ou à l'un de ces dossiers.

des sénateurs n'appartenant à aucun groupe. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est la question que se posent des millions de Français après avoir appris que quinze membres de votre gouvernement étaient candidats aux élections régionales ou départementales. Alors que la France est plongée dans une crise sanitaire, économique et sécuritaire inédite dans l'histoire, vos ministres n'ont manifestement rien de mieux à faire que d'aller distribuer des tracts ou coller des affiches, avec Rolex, ou Bréguet, et boutons de manchette aux poignets. Le ministre

Mme Schiappa est aussi candidate, mais comme sa seule activité est de faire des tweets, personne ne verra la différence. Le ministre de la santé a même affirmé qu'il irait coller des affiches de Renaud Muselier dans ma région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pendant ce temps, des Français souffrent, sont au chômage, dorment dans la rue ou dans leur voiture, se font agresser, y compris des maires de petites communes. Pendant que vous faites campagne et que vous découvrez le pays- c'est déjà cela ... -, des restaurateurs, des hôteliers des cafetiers se battent tous les jours pour survivre. Pendant ce temps, les jardins de l'Élysée se transforment en théâtre de Guignol ; c'est non plus le, mais le ... Charles, François, réveillez-vous : ils sont devenus fous

la proposition de loi que je présente au nom du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires comprend une mesure immédiate de lutte contre l'aggravation de la pauvreté résultant de la crise sanitaire, ainsi que son financement solidaire. Le constat social est sans appel et s'aggrave de jour en jour : selon les associations nationales de solidarité du collectif Alerte,

Bien avant que les statistiques de l'Insee ne mesurent le recul du niveau de vie des plus précaires, ces acteurs, au plus près du terrain, alertaient sur la dégradation de la situation sociale au travers d'indicateurs probants explosion du recours à l'aide alimentaire et arrivée massive de nouveaux publics, dont des jeunes, des étudiants et des indépendants. Quant aux départements, ils enregistraient une augmentation rapide des demandes d'allocation du revenu de C'est à ce contexte plus qu'alarmant que nous souhaitons apporter une première réponse. Le retour du creusement des inégalités a certes précédé la crise et trouve sa source dans les mesures fiscales ou de dérégulation que nous avons dénoncées en leur temps et auxquelles nous continuerons d'apporter des réponses structurelles dans de prochaines propositions de loi, afin de renouer avec le progrès social. Mais, pour les plus vulnérables, le surcroît de difficultés dans ce contexte de pandémie est dû à l'insuffisance des mesures d'accompagnement gouvernementales. Privés d'actions publiques fortes de soutien, ces ménages sont passés en quelques mois d'une situation plus que fragile à une situation dans laquelle ils ne parvenaient plus du tout à faire face à leurs besoins fondamentaux, voire vitaux. C'est ce constat partagé par les acteurs de la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion qui nous invite à adopter sans attendre des mesures d'urgence propres à la situation de crise qui nous conduit à formuler cette proposition d'une aide forfaitaire mensuelle, ciblée sur le public le plus défavorisé, rapidement opérationnelle et automatisable. Nous avons alors délimité le périmètre le plus pertinent d'application de la mesure. La capacité à faire face à la situation de crise, notamment de confinement, s'est révélée dans le mouvement de croissance du patrimoine financier net dû à l'épargne supplémentaire,

Sans grande surprise, sur près de 200 milliards d'euros d'épargne supplémentaire, la Banque de France et différents organismes d'analyse convergent pour estimer que les 20 % de ménages aux revenus les plus faibles ont désépargné ou se sont endettés à hauteur de 2 milliards d'euros pour la seule première période de confinement. Inversement, quelque 70 % de l'épargne supplémentaire étaient concentrés chez les 20 % de ménages aux plus hauts revenus. Par ailleurs, la Fondation Abbé Pierre, qui a analysé les arbitrages de dépenses des ménages pauvres lors de la crise financière de 2008, nous enseigne en cas de baisse de ressources, comme aujourd'hui, ces ménages privilégient le paiement du loyer, ce qui augmente le taux d'effort. Face à la baisse du reste à vivre, réduit à une poignée d'euros par jour et par personne- on parle de 9 euros rationnent les autres dépenses, alimentaires et de soins notamment. Les impayés de loyer surviennent plus tard, quand la baisse des ressources perdure et que l'épargne est épuisée.

La moitié des économies budgétaires induites par ces réformes ayant été réalisée sur le dos des 20 % les plus pauvres, la moitié de notre aide d'urgence ira également vers la même population et le reste sur les déciles proches. Enfin, de toutes les prestations, ce sont les APL qui ont le plus fort impact social et l'effet redistributif le plus puissant : elles réduisent de près de 8 points l'intensité de la pauvreté. Si les APL sont le support, c'est parce qu'elles délimitent le public prioritaire dans le cadre d'une mesure d'urgence de soutien au pouvoir d'achat à destination des plus touchés par la crise. Nous vous proposons donc de voter l'article 1, qui prévoit une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros par mois à compter de la promulgation de la loi et jusqu'à trois mois après la fin de l'état d'urgence. Concernant la compensation financière de cette dépense étatique, nous proposons de décaler d'un an, comme cela s'est déjà produit, le dispositif de la deuxième tranche d'exonération de la taxe d'habitation des 20 % de ménages les plus aisés,

les plus aisés, dans un contexte où ceux-ci ont constitué des niveaux inégalés d'épargne en un temps très court. Notons en effet

Ce cadeau fiscal, qui a le même effet qu'une dépense sur l'équilibre budgétaire de l'État et qui a été justifié au nom d'un principe d'égalité désincarné, se révèle de fait particulièrement inéquitable. s'agit cependant pas de revenir sur cette baisse initialement pensée pour les classes moyennes, dès à présent exonérées, mais de la décaler d'un an, dans le contexte exceptionnel de la crise, afin de préserver des marges de manoeuvre financières à l'État pour assurer plus fortement son rôle de protection des plus vulnérables. C'est l'objet de l'article 2. Mes chers collègues, l'accroissement des inégalités de revenus et de patrimoine, démultipliées en période de crise, reste, quel que soit le contexte économique, incompatible avec la lutte contre la pauvreté et contre le recul du niveau de vie des plus précaires. L'urgence sociale nous invite à des mesures immédiates, justes et solidaires. Je vous demande d'adopter l'une d'elles en votant cette proposition de loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise comprend deux articles, le second étant présenté comme une compensation des conséquences financières du premier. L'article 1 prévoit le versement d'un complément de 100 euros par mois aux bénéficiaires des aides personnelles au logement. Cette mesure s'appliquerait jusqu'à trois mois après la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire jusqu'à la fin août de cette année si l'état d'urgence n'est pas prorogé au-delà du 1 juin. Cette mesure est rattachée par ses modalités aux aides au logement, ce qui faciliterait certainement sa mise en oeuvre, mais elle est en fait d'une nature très différente. elle ne dépend pas du niveau du loyer, des ressources, du patrimoine ou même du nombre de personnes composant le ménage : l'aide serait identique pour une famille nombreuse sans ressources, qui bénéficie en conséquence d'une APL relativement élevée, et pour une personne seule à revenu plus élevé, pour laquelle le niveau de l'APL est réduit. Il s'agirait donc d'une aide sociale générale, sans véritable lien avec les dépenses de logement, mais dotée d'un effet de seuil considérable, puisqu'une légère différence de revenus suffirait pour qu'un ménage bénéficie, ou non, de l'intégralité de l'aide de 100 euros. Le coût est facile à estimer le nombre des bénéficiaires des aides personnelles au logement étant d'environ 6,6 millions d'euros, la mesure représenterait une dépense de l'ordre de 660 millions d'euros par mois, ou 2 milliards d'euros pour trois mois. Pour mémoire, le montant total des aides personnelles au logement a été de 17 milliards d'euros en 2020, dont 13,9 milliards d'euros à la charge de l'État. L'article 1 gage cette dépense sur les recettes provenant du report de la mise en oeuvre de la taxe d'habitation à l'article 2, mais ces recettes seront nulles en 2021. En pratique, c'est donc une taxe additionnelle aux droits sur le tabac qui devrait être créée. dont la création repose sur le souhait légitime d'aider les ménages à revenus modestes pendant la crise sanitaire, me semble mal adaptée à la diversité de leur situation, ainsi qu'à leur exposition réelle aux effets de la crise, qui dépend d'autres facteurs, tels que le secteur économique d'activité ou le type de contrat de travail. La commission des finances n'a donc pas adopté cet article. L'article 2 de la proposition de loi a pour objet de modifier la trajectoire de suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour ce qui concerne, plus particulièrement, l'allègement en faveur des « 20 % de ménages aisés La mesure a un double objectif d'après les auteurs de la proposition de loi. Tout d'abord, elle vise à dégager des ressources pour assurer le financement des aides proposées à l'article 1. Ensuite, elle prévoit d'organiser une contribution plus importante des ménages que l'exposé des motifs qualifie de « privilégiés ». Mes chers collègues, je me permettrai de vous présenter un bref rappel des grandes lignes de la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales, avant de vous expliquer plus précisément le contenu de la À l'occasion de la loi de finances pour 2018, le Parlement a adopté, comme vous le savez, un dégrèvement progressif de la taxe d'habitation sur les résidences principales en faveur des « 80 % de ménages les moins aisés Ainsi, en 2020, les ménages concernés ont bénéficié d'un dégrèvement intégral de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Dans la loi de finances pour 2020, le Parlement a voté la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales à compter de 2023. Cette réforme comporte plusieurs volets. En premier lieu, le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences principales est transformé en exonération. En deuxième lieu, les « 20 % de ménages aisés restant redevables de la taxe dans le dispositif introduit en 2018, bénéficieront d'une exonération progressive en 2021

En troisième lieu, à compter de 2021, le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales est intégralement reversé à l'État. Enfin, la réforme prévoit que les collectivités locales bénéficient de ressources de substitution, au travers, vous le savez, de la redescente de la part départementale de la taxe foncière ou de l'affectation d'une fraction de TVA. La commission des finances et le Sénat ont largement discuté et débattu de cette réforme, que nous jugions, je le rappelle, critiquable sur de nombreux points. En particulier, nous avions considéré que l'impact sur les collectivités locales de la mise en oeuvre de ce nouveau modèle de financement n'était pas suffisamment évalué. Le Sénat avait donc, sur l'initiative de la commission des finances, voté une série d'amendements tendant à décaler d'un an la mise en oeuvre du nouveau schéma de financement des collectivités locales. Je me permets d'insister sur ce dernier point ce que le Sénat a voté, c'est un décalage d'un an de la redescente de la taxe foncière et de l'affectation de TVA aux établissements À aucun moment, le Sénat n'a remis en question par son vote le principe ou la trajectoire d'allègement en faveur des 20 % de ménages restant redevables de l'impôt. Celle-ci s'impose pour des motifs constitutionnels, comme l'analysait fort bien le rapport Richard-Bur de 2017. J'en viens au contenu de l'article 2 de la proposition de loi. Il prévoit que l'exonération à 65 % de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui doit s'appliquer en 2022 au profit des 20 % des ménages restant redevables de l'impôt, soit limitée à 30 %. L'exonération à 65 % ne s'appliquerait qu'en 2023, et la taxe ne serait supprimée, d'abord, je rappelle que ces propositions sont absolument sans incidence pour les collectivités locales, qui n'y gagneront ou n'y perdront rien. En effet, le nouveau schéma de financement des collectivités locales est déjà en vigueur : c'est donc l'État qui perçoit actuellement la taxe d'habitation sur les résidences principales. Ne voyons donc pas là, mes chers collègues, une occasion de refaire le match de la réforme

la mesure a pour objet d'engendrer une recette supplémentaire pour l'État de l'ordre de 2,6 milliards d'euros en 2022, afin de financer le coût des aides prévues à l'article 1. Par cohérence avec la proposition de rejet de cet article que j'ai déjà évoqué, je considère que le dispositif de l'article 2 ne se justifie plus. Deuxièmement, la mesure vise, selon ses auteurs, à renforcer la justice fiscale en organisant une plus forte participation des ménages « favorisés ». Ce terme est, me semble-t-il, loin d'être adéquat. Certes, les ménages encore redevables de la taxe d'habitation disposent, par définition, des 20 % de revenus les plus importants. Néanmoins, il faut rappeler que cette présentation ne rend pas compte du fait que les seuils retenus sont en réalité assez faibles et que l'on peut être, dans une pièce comptant dix personnes, parmi les deux qui gagnent le mieux leur vie sans pour autant être riche. Par exemple, un couple sans enfant figure parmi les 20 % de ménages aisés dès lors que le revenu mensuel de chacun des conjoints excède 1 749 euros après impôts. Pour un couple avec deux enfants, ce montant est de 2 256 euros. Il s'agit pour moi non pas de nier le fait qu'une part importante de nos concitoyens perçoit des revenus inférieurs à ceux que je viens de citer, mais plutôt de rappeler que l'on ne peut pas vraiment dire que les ménages visés par la mesure proposée sont des « privilégiés ». En troisième et dernier lieu, j'indiquerai que revenir sur le niveau de l'exonération applicable en 2022 serait un mauvais signal. Ce serait un mauvais signal pour le soutien à la relance, car cela réduirait le pouvoir d'achat des ménages qui s'attendaient à bénéficier de cette mesure. Ce serait un mauvais signal pour la prévisibilité de la loi de fiscale également, alors que celle-ci constitue un élément de confiance important. Pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées, la commission des finances n'a adopté aucun des deux articles de la proposition de loi et vous propose donc de rejeter celle-ci.

nous nous entendons sur le constat et les problèmes. En premier lieu, nous partageons évidemment le constat que vous avez dressé, madame la sénatrice : la crise sanitaire a incontestablement aggravé les inégalités. Par de nombreux aspects, la crise du covid affecte plus durement les ménages en bas de l'échelle de revenus, pour différentes raisons. Ces ménages sont plus nombreux à travailler dans des secteurs particulièrement pénalisés par la crise, comme la restauration ou les transports.

d'actualité au Gouvernement- pardonnez-moi cette redondance ! -, une étude du Trésor de fin 2020 montrait que les deux tiers des bénéficiaires des aides débloquées pour les ménages afin de faire face à la crise figuraient parmi les 20 % des Français les moins riches. signifie certainement pas que la question est réglée, mais on peut au moins dire que la réponse a été rapide, juste et solidaire. En l'état, la bonne nouvelle est que nous faisons le même constat et que nous faisons mieux que partager la solution : nous l'appliquons. Pour autant, si d'autres moyens peuvent être fort légitimement envisagés pour amplifier l'aide à nos concitoyens les plus modestes, nous divergeons clairement sur la nature de ces moyens. L'article 1 de la proposition de loi prévoit le versement d'une aide de 100 euros par mois aux bénéficiaires des aides au logement, à compter de la promulgation de la loi et jusqu'à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, prévue le 1 juin Cette proposition présente plusieurs limites, déjà évoquées par M. le rapporteur. En premier lieu, le montant prévu n'est pas nécessairement proportionné ou adapté aux besoins des foyers ; en particulier, il ne dépend pas de la configuration familiale.

le versement d'une aide exceptionnelle ciblée vers les bénéficiaires d'une prestation suscite ou renforce des effets de seuil importants, qui, s'ils peuvent être raisonnables dans le cas d'un versement ponctuel, seraient amplifiés dans le cas de versements répétés.

Pour rappel, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes et de façon bornée dans le temps- de 2020 à 2023 -, de la taxe d'habitation sur l'habitation principale. principale. Or- ce n'est pas à vous que je le rappellerai -c'est un principe constitutionnel qui a incité le Gouvernement à amplifier cet engagement du Président de la République, dont la proposition initiale ne visait pas, c'est vrai, les 20 % des ménages les plus aisés. dans sa décision sur le projet de loi de finances pour 2018, le Conseil constitutionnel a clairement rappelé qu'il se réservait la possibilité de réexaminer cette disposition au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, en fonction notamment de la façon dont serait traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation. De même, le Conseil d'État estime qu'un dispositif consistant en un impôt national calculé à partir d'assiettes localement définies et de taux déterminés par les collectivités locales méconnaîtrait, s'il était pérenne, les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, mais pourrait être admis à titre transitoire « pour une durée courte, par exemple d'un ou deux ans ». Ainsi, le décalage d'un an de l'échéancier de suppression de la taxe d'habitation pourrait être perçu comme un renoncement à la réforme, ce que nous ne souhaitons pas, et présenterait en outre un fort risque d'inconstitutionnalité, ce que nous ne souhaitons pas davantage.

La diminution de la pauvreté demeure pour nous une boussole, et c'est avec cette boussole que nous avons déterminé le chemin que nous suivons depuis le début de la crise. Rappelons tout d'abord le formidable amortisseur de la baisse des revenus du travail qu'ont représenté la mise en place de l'activité partielle, celle du fonds de solidarité et l'extension des indemnités journalières.

laquelle a été étendue également aux familles bénéficiaires des aides au logement, ce qui représente près de 4,1 millions de bénéficiaires. Par ailleurs, les étudiants en difficulté et les jeunes précaires de moins de 25 ans ont reçu une aide de 200 euros en juin 2020 ; cela a concerné environ 800 000 bénéficiaires.

l'aide exceptionnelle aux bénéficiaires du RSA et des aides au logement a été renouvelée en novembre 2020 et une aide de 150 euros a également été versée aux étudiants boursiers et aux jeunes non étudiants percevant les allocations logement. Par ailleurs,

chargé du suivi et de l'évaluation des mesures de soutien, nous a indiqué que, contre vents et marées, le pouvoir d'achat s'était maintenu à un niveau stable en 2020. Bien entendu, il faut manier les agrégats avec précaution et discernement néanmoins, les mesures de soutien mises en place par le Gouvernement ont joué leur rôle, car le choc de la crise sur les revenus a été absorbé à 65 % par les administrations publiques, à 31 % par les entreprises et à 4 % seulement par les ménages. Sur la même période, l'emploi n'a reculé que de 1,6 %, en raison d'un dispositif d'activité partielle d'une ampleur inédite. Cette résilience est inattendue, mais elle ne doit pas pour autant nous faire oublier que la crise a touché plus durement les ménages les plus modestes. C'est cette question qui anime nos collègues qui sont à l'origine de cette proposition de loi, mais c'est également, reconnaissons-le, un sujet qui nous rassemble très largement sur les différentes travées. Cette question a tout pour nous rassembler.

les écueils de cette proposition de loi ont été également été relevés par les différents groupes qui se sont exprimés. Je ne reviendrai pas en détail sur les objections de fond évoquées par M. le rapporteur. Je me contenterai de rappeler que l'article 1 prévoit une aide forfaitaire pour tous les bénéficiaires des aides au logement, indépendamment du niveau de loyer, des ressources, du patrimoine ou de la composition du foyer une mesure particulièrement large, insuffisamment ciblée et qui souffre d'importants effets de seuil. Non seulement l'article 2 ne permettra pas de financer la mesure, en raison de la non-concordance des dates, mais il va à contre-courant du vote du Parlement, qui s'était prononcé sur la trajectoire de suppression de la taxe d'habitation en loi de finances initiale, et à rebours de l'engagement du Gouvernement de ne pas alourdir la charge fiscale en période de reprise. Cela dit, parce que la question que pose cette proposition de loi mérite toute notre attention,

Ces crédits ont permis de financer les aides exceptionnelles de solidarité annoncées par le Président de la République ainsi que par le Premier ministre, au mois d'octobre 2020. Ces mesures comprenaient non seulement un versement de 150 euros pour les foyers bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite, mais également une aide de 100 euros par enfant à charge pour les foyers percevant des APL, ainsi que, enfin, une aide de 150 euros pour les jeunes de moins de 25 ans, apprentis, étudiants salariés ou non-étudiants, qui perçoivent une aide personnelle au logement. donc ici, mes chers collègues, trois exemples de mesures efficientes, équilibrées et qui viennent spécifiquement en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Notre secrétaire d'État nous confirme que ces dispositifs se poursuivront, en étant adaptés autant que nécessaire. J'en conviens, on n'en fera jamais trop pour accompagner les Français en difficulté. Aussi, vous pourrez toujours compter sur le groupe RDPI pour travailler à des propositions concrètes et mesurées. Toutefois, dans un souci de cohérence avec la politique gouvernementale

Elle prévoit en outre de modifier le calendrier de l'exonération de la taxe d'habitation pour financer cette mesure. Le dispositif envisagé consiste à verser aux bénéficiaires des aides personnalisées au logement un complément d'un montant de 100 euros par mois, jusqu'à trois mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

L'article 1 instaure le complément de 100 euros, soit une augmentation de 65 % à 100 % du montant des APL pour les étudiants y ayant droit et de près de 50 % du montant moyen des APL, soit 225 euros, pour 6,6 millions de foyers concernés. Cette aide massive s'appliquerait dès la promulgation du texte, en urgence. L'article 2, quant à lui, modifie l'article 16 de la loi de finances pour 2020, portant dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale des 20 % de ménages les plus aisés : il en reporte la deuxième étape de 2022 à 2023 et la suppression définitive de la taxe Si- je tiens à le rappeler -la suppression de la taxe d'habitation est une erreur à la fois financière et démocratique, il ne me semble pas judicieux de revenir sur le calendrier établi. Les auteurs de ce texte ont également voulu apporter une réponse politique à la baisse de 5 euros des APL, décidée par le Gouvernement en début de mandat, mandat, et à la réforme actuelle de ces aides, insatisfaisante, j'en conviens, en particulier pour ce qui concerne l'accession à la propriété. Social Européen approuve la volonté affichée de lutter contre l'aggravation des inégalités dans la crise, la solution choisie ne semble pas vraiment adaptée aux besoins réels de la population.

Les inégalités patrimoniales étaient encore plus fortes, et 9,3 millions de personnes avaient un revenu inférieur au seuil de pauvreté. En 2020, un million de personnes supplémentaires se retrouvent en situation de pauvreté, soit plus de 10 millions de nos concitoyens.

Or les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont confrontées à des arbitrages insolubles au quotidien : payer les factures ou manger, payer les factures ou se loger, se vêtir, chauffer son logement ou encore se soigner, payer l'assurance, le transport, les impôts ou les crédits en cours. Le reste à vivre diminue comme peau de chagrin, en raison de la part prépondérante des dépenses de logement, le loyer représentant en moyenne 36 % des dépenses des ménages précaires. Dans ce texte, rien ne vient garantir que les 7 milliards d'euros que coûterait cette disposition seraient véritablement utiles pour lutter contre les inégalités, et il y aurait, à coup sûr, un effet de seuil considérable entre les bénéficiaires de cette mesure et les autres. C'est

notamment en raison des minima sociaux, les bénéficiaires d'aides au logement pauvres sont aussi pauvres que l'ensemble des personnes pauvres ». Si la tournure de phrase peut paraître quelque peu déconcertante, elle a au moins le mérite d'insister sur le niveau de précarité des allocataires des APL.

nous nous étions joints à ce constat -n'était pas une réponse adaptée pour les plus précaires. Ainsi, lorsque, selon la version du Gouvernement, une famille au RSA de trois enfants percevait 450 euros pour le seul versement de novembre, elle touche 50 euros de plus que ce à quoi elle pourrait prétendre avec l'aide totale de nos collègues écologistes. insuffisante, ensuite, car l'un des objectifs de la proposition serait de remédier à la précarité manifeste et d'ampleur dans laquelle a basculé la jeunesse. Or, des 2,9 millions d'allocataires des APL, seulement 15 % ont moins de 29 ans et seulement 5 % sont étudiants, ce qui représente 133 000 allocataires.

et écologiste avait proposé de revaloriser les bourses et les minima sociaux, d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, de compenser à 100 % le dispositif d'activité partielle pour les travailleurs modestes. Il y aurait là de véritables réponses solidaires face à la crise sanitaire. Quant au logement, le groupe CRCE a fait adopter, dans cet hémicycle, voilà quelque temps, une proposition de loi tendant à revenir sur le délai de carence et la réindexation des APL. Ces mesures auraient permis une revalorisation pérenne des aides, au plus près des réalités économiques de ceux qui en ont besoin. Nous voterons en faveur de cette aide de 100 euros par mois, limitée aux trois ou quatre prochains mois, mais nous nous opposerons à son financement, prévu à l'article 2. En effet, le simple décalage d'un an de l'exonération de taxe d'habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés ne constitue ni une réponse face à la crise ni une mesure de justice sociale. Nous avions mené ardemment le combat contre cette réforme injuste, qui pèse sur les finances locales et profite aux plus aisés. Prenons l'exemple de Maubeuge : dans cette ville, un tiers des foyers ne payaient pas la taxe d'habitation ces ménages la financent indirectement, l'acquittement la TVA, qui s'applique à tous. Pourquoi transférer ainsi la charge sur les foyers précaires ?

la pandémie de la covid-19 a provoqué une multitude de mutations économiques, sociales et financières, dont un accroissement des inégalités. Face à ce constat, la présente proposition de loi vise- cela a été indiqué -à apporter une réponse solidaire et juste face à la crise. Si l'objectif affiché repose sur un constat partagé, les différentes dispositions du texte ne semblent pourtant en adéquation ni avec la volonté politique originelle ni avec le contexte socioéconomique actuel. L'article 1 de la proposition de loi prévoit le versement d'un complément de 100 euros par mois aux bénéficiaires des aides personnelles au logement jusqu'à trois mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cette disposition présente plusieurs limites. Tout d'abord, le caractère universel de cette augmentation ne permettrait pas de cibler les populations les plus fragiles financièrement ; la mesure ne prévoit aucune prise en compte de la diversité des situations. Des critères objectifs tels que le taux d'effort permettraient, par exemple, de mieux épouser les réalités individuelles. Il existera alors un réel effet de seuil : une légère différence de revenus suffira pour qu'un ménage bénéficie, ou non, de l'intégralité de l'aide de 100 euros. Ensuite, cette augmentation généralisée des aides personnelles au logement tendrait à renforcer les inégalités inhérentes au calcul de ces dernières. Dans son rapport annuel d'activité pour l'année 2019, la Cour des comptes insiste sur le caractère inégalitaire des APL, en raison d'un mode de calcul toujours plus complexe. En ce sens, la disposition prévue à l'article 1 contribuerait à renforcer une dynamique déjà inégalitaire, au lieu de la corriger. Par ailleurs, le fait d'accroître le montant des APL se traduirait également par un coût non négligeable pour les finances publiques. finances publiques. La mesure représenterait une dépense de l'ordre de 660 millions d'euros par mois, soit de près de 2 milliards d'euros pour trois mois. Pour rappel, le montant total des aides personnelles au logement s'est élevé à 17 milliards d'euros en 2020. Étant donné les effets limités de cette disposition, cela ne justifie pas un tel effort financier de la part de l'État et, indirectement, de la part des contribuables français. En outre, l'article 1 de la présente prévoit une aide générale et automatique ne reposant sur aucune équité sociale. Cette mesure se révèle déconnectée de la diversité des situations et coûteuse pour les finances de l'État.

suppression. Plusieurs points de vigilance doivent être soulignés. Premièrement, la mesure susciterait une recette supplémentaire, pour l'État, de l'ordre de 2,6 milliards d'euros en 2022, afin de financer le coût des aides prévues à l'article 1. 1. Le raisonnement que je vous ai exposé en défaveur de cet article rend naturellement le maintien de l'article 2 totalement incohérent. Deuxièmement, cet article s'attaque à une réforme déjà engagée. Il me paraît peu pertinent de raviver les débats autour de cette réforme structurelle, en y appliquant une modification substantielle de calendrier, modification qui aurait un effet direct sur la prévisibilité de loi fiscale et sur la pression fiscale d'une partie des contribuables. l'argument politique consistant à mettre à contribution les 20 % des revenus les plus aisés- les « plus privilégiés », pour citer l'exposé des motifs de la proposition de loi -, en maintenant la taxe d'habitation pour ces derniers, ne semble pas se traduire dans le texte présenté. Par exemple, un couple sans enfant figure parmi les 20 % de ménages aisés dès lors que le revenu mensuel de chacun des conjoints excède 1 749 euros après impôts l'existence de revenus dits « aisés » ne suffit pas à caractériser la richesse d'un ménage. Il s'agit donc non d'un moyen de favoriser la justice sociale, mais du report d'un allègement fiscal pour une partie des classes moyennes. Enfin, dans la mesure où la reprise économique reste nécessaire, après la période de la covid, le fait de maintenir cette taxe représenterait un frein pour la consommation.

les dispositions prévues dans le texte supposent le déploiement d'importants moyens financiers pour des effets très limités. Ainsi, pour reprendre les mots du rapporteur général, lors de l'examen en commission, « cette proposition de loi apporte une réponse inadaptée, inappropriée,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires de nous permettre de nous pencher à nouveau sur les conséquences sociales de la pandémie et de porter une proposition de loi utile pour les personnes qui sont le plus en souffrance.

si l'on peut tout à fait admettre que, en période de croissance, une partie des recettes nouvelles permette la diminution des taux d'imposition tant des ménages que des entreprises, comment comprendre

est pleinement justifié. Pour tout dire, je le trouve même modéré ; pour ma part, je considère qu'aucune baisse d'impôt n'a de sens tant que l'on n'aura pas retrouvé le niveau de PIB que l'on aurait dû avoir sans la crise,

de la taxe sur les dividendes, et après la création de la, un énième cadeau offert aux plus aisés, alors que le pays traverse une crise sans précédent. Comme si cela ne suffisait pas, le Gouvernement se prive annuellement de 10 milliards d'euros d'impôts de production, au nom de la relance, alors que cette demande du monde économique est aussi vieille qu'injustifiée dans la période

Parallèlement, du rapport Arthuis sur l'avenir des finances publiques au nouveau programme de stabilité, on ne jure plus que par la réduction de la dépense publique, au nom de la stabilisation de la dette. Cela ne manque pas de sel Lors de la crise financière de 2008, le Gouvernement avait renoncé à sa promesse de diminuer les prélèvements obligatoires, afin de préserver les recettes de l'État. De votre côté, madame la secrétaire d'État, vous refusez d'intégrer les conséquences de la pandémie dans votre logiciel.

Oui, madame la secrétaire d'État, nous pouvons avoir une réflexion sur notre dépense publique et sur notre fiscalité ; oui, en période de croissance économique, tout peut se discuter. Mais, en période de crise, il y a malheureusement bien d'autres priorités. Le déficit à financer pour 2020 s'élève à 206 milliards d'euros. Madame la secrétaire d'État, vous désirez atteindre 3 % de déficit public en 2027 ; pour y parvenir, il faudrait réaliser 65 milliards d'euros d'économies. À l'heure actuelle, peu de mesures concrètes sont annoncées, alors que cet effort est considérable. J'ai toutefois ma petite idée- je vous en parlerai -quant aux directions que vous prendrez En temps de crise, l'État-providence doit jouer pleinement son rôle, ... Il l'a joué ! ... notamment en protégeant les Français les plus modestes des aléas économiques. C'est notre ambition, et cela peut passer par la revalorisation des APL le temps d'une crise sanitaire, comme le propose le groupe GEST, afin de cibler les familles les plus en difficulté. Depuis le début de la crise, les groupes de gauche de la Haute Assemblée ont été force de proposition pour faire face

utile à la crise socioéconomique. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera, sans surprise, mais avec conviction, pour cette proposition de loi. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « ce ne sont [ ...] pas les faits en eux-mêmes qui frappent l'imagination populaire, mais bien la façon dont ils sont répartis et présentés. Il faut que par leur condensation, si je puis m'exprimer ainsi, ils produisent une image saisissante qui remplisse et obsède l'esprit. Qui connaît l'art d'impressionner l'imagination des foules connaît aussi l'art de les gouverner Depuis que Gustave Le Bon a publié sa, on sait qu'il suffit de répéter un mensonge un très grand nombre de fois pour qu'il paraisse la réalité. En France, les chiffres d'Oxfam et compagnie tentent de faire naître en nos esprits cartésiens l'image d'une France trop inégalitaire. Or il suffit d'analyser les principaux indicateurs de répartition des richesses pour comprendre que, même s'il y a de nombreux problèmes d'inégalités dans notre pays, la France est très loin de tomber dans cette caricature. Le plus connu d'entre eux est le coefficient de Gini, qui varie de 0 à 1 et situe un pays entre deux positions extrêmes : 0, dans le cas où tous les citoyens possèdent exactement la même chose ; 1, dans le cas où un citoyen possède toutes les richesses et les autres aucune.

Bien sûr, on trouve toujours des spécialistes des inégalités pour expliquer que cet indicateur synthétique masque, en fait, de grandes disparités, notamment entre les plus riches et les plus pauvres. là encore, le cas de la France ne correspond pas à la critique. Ainsi, si on évalue le rapport interdécile, qui compare ce que touchent en moyenne les 10 % les plus favorisés et les 10 % les moins favorisés, la France fait encore mieux. Avant la crise, les 10 % les plus favorisés touchaient environ 7 fois plus que les 10 % les moins favorisés. L'exposé des motifs de la proposition de loi rappelle ce chiffre.

voulez ? La France est tout sauf un pays qui laisse les inégalités se creuser, comme on laisserait les gens mourir de faim. C'est faux ! Avec une dépense publique qui a atteint, pendant la crise, la barre symbolique de 60

mais toutes les mesures d'urgence sont encore activées. Les millions de chômeurs qui arrivaient en fin de droits pendant la crise ont vu leurs allocations prolongées ; l'État a financé tous les salaires des travailleurs qui risquaient d'être licenciés le Gouvernement a augmenté le salaire des soignants- c'est bien normal -et baissé les impôts des entreprises. Apparemment, c'est encore trop peu. La véritable urgence, aujourd'hui, c'est d'inventer de nouveaux modèles économiques pour rembourser la dette astronomique que nous avons contractée au cours de la crise. Il faudra, pour cela, investir massivement dans la transition écologique et développer de nouvelles verticales d'innovation et de nouvelles industries susceptibles de créer de l'emploi.

les plus pauvres, ceux qui ont pioché dans leurs bas de laine ou qui se sont endettés de 2 milliards d'euros pendant la première phase de cette crise. Dans le même temps, les 10 % les plus riches, eux, augmentaient leur bas de laine de 25 milliards d'euros Ceux qui ont gonflé les files d'attente devant les associations d'aide alimentaire sont là, même si Mme Paoli-Gagin ne les voit pas. Ce sont des jeunes, des familles monoparentales, des Français qui vivent dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales éloignées,

Je voudrais vous parler de ceux qui ont remis à plus tard non pas leur voyage, leur sortie au restaurant ou leur soirée au théâtre, mais leur rendez-vous chez le médecin, le dentiste ou l'ophtalmologue, ceux qui n'ont pas pris de mutuelle ou ceux qui ont pioché dans leurs économies pour payer leur loyer.

payer l'endettement de l'Unédic, lié notamment au chômage partiel, en diminuant l'assurance chômage pour les plus précaires. Nous vous exhortons également à cesser de mépriser sans cesse les plus pauvres, dans vos discours et dans vos actes.

les personnes seules, les retraités, les personnes seules avec enfants, les étudiants, ainsi que beaucoup d'autres catégories. Des constats sont dressés, depuis de très nombreuses années, sur l'existence de situations particulièrement difficiles,

Comme l'a indiqué notre rapporteur Charles Guené au sujet des deux articles de cette proposition de loi, il est important de rappeler le coût budgétaire des aides personnelles au logement, qui s'élève,

L'article 1 de proposition de loi prévoit un complément d'aide au logement de 100 euros par mois aux personnes et ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement. La commission des finances indique que le dispositif est coûteux, s'il s'applique pour une durée limitée jusqu'à la fin août 2021, sauf prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Le coût de cette mesure est estimé à 660 millions d'euros par mois, sur un coût global de 2 milliards d'euros. En outre, ce dispositif n'est pas proportionné

culture. L'article 2 vise un report d'un an de la trajectoire d'exonération progressive des ménages demeurant redevables de la taxe d'habitation au titre des résidences principales. Le rapporteur a rappelé le droit existant : exonération progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales applicable jusqu'à la suppression en 2023 de cet impôt dont le produit résiduel est aujourd'hui perçu par l'État, alors que les collectivités locales bénéficient de ressources de substitution.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous faisons, hélas, le même constat que nos collègues du groupe écologiste. Les inégalités, la pauvreté et la précarité se sont singulièrement aggravées depuis le début de la crise sanitaire. précarité risque de s'accroître encore plus lorsque les diverses mesures de soutien aux entreprises prendront fin. Nous approuvons la démarche de nos collègues d'y apporter une première réponse, centrée sur le logement. La discussion de cette proposition de loi est pour nous l'occasion de vous interpeller, madame la secrétaire d'État, sur la politique du logement menée par le Gouvernement depuis 2017 : baisse de 5 euros, puis désindexation, puis contemporanéisation des Le logement fait indiscutablement partie des politiques publiques sacrifiées depuis 2017. Même pendant la crise sanitaire, vous n'avez eu de cesse de le considérer comme une variable d'ajustement budgétaire. Si les récentes annonces du Premier ministre en la matière semblent aller dans le bon sens, nous attendons de votre part une réelle prise de conscience, qui se traduise par une politique du logement beaucoup plus ambitieuse. L'augmentation de 100 euros des APL, proposée par nos collègues du groupe écologiste, est une réponse d'urgence, qui permettrait de soutenir immédiatement plus de 6 millions de foyers et 13 millions de nos compatriotes. Bien sûr, tout est perfectible, et d'aucuns trouveront le montant trop ou pas assez élevé, ou encore pas proportionné. Il s'agit là d'un dispositif temporaire, qui doit permettre l'élaboration des mesures adaptées à la diversité des situations. En ce sens, et en toute logique, cela ne devrait en aucun cas invalider en aucun cas invalider le vote de cet article, quitte à ce qu'il soit amendé le cas échéant. Le report d'un an de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés permettrait de financer cette mesure solidairement. Nous avions d'ailleurs nous-mêmes proposé de décaler l'entrée en vigueur de la réforme de la taxe d'habitation d'un an, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, afin de financer de nouvelles mesures de solidarité pour soutenir les ménages les plus modestes, compte tenu de l'urgence sociale. Le Gouvernement avait alors rejeté notre proposition. En cette période de crise sanitaire, mais aussi économique et sociale, il nous semble en effet plus que jamais utile et sain d'allier justice sociale et justice fiscale et de prendre des mesures redistributives en direction de nos compatriotes les plus en difficulté.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

la présidente. Acte est donné du retrait de la proposition de loi par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires de l'ordre du jour de son espace réservé.

les pandémies questionnent à chaque fois notre rapport à l'animal, qu'il soit sauvage ou domestique, ainsi que notre modèle agricole et notre système de santé. Ce n'est pas sans fierté que je vous présente ce jour, au nom du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, une proposition de loi

J'ajouterai, à titre liminaire, que ce texte a reçu le soutien de nombreuses associations de défense des droits des animaux, mais aussi l'assentiment de sénateurs et sénatrices membres de six groupes politiques différents, que je tiens à remercier. C'est dire la résonance globale de ce sujet dans notre société, au-delà des clivages partisans. L'élevage intensif est vivement critiqué relativement au bien-être animal et à la qualité de la viande, ainsi qu'aux conditions de travail des professionnels et à son modèle.

Ces animaux subissent dans des « fermes-usines » des traitements cruels et parfois intolérables. Ils se trouvent confinés, sans accès à des espaces de plein air et souvent dans des cages, ce qui entraîne chez eux des troubles comportementaux extrêmes. Les élevages précités asphyxient en outre les productions locales, qui ont vu leur nombre baisser drastiquement ces dernières années. Ce sont alors les agriculteurs eux-mêmes qui pâtissent grandement de prix non rémunérateurs, associés à des conditions de travail difficiles, contribuant lourdement au mal-être du monde agricole. C'est pourquoi, à des fins de promotion d'un modèle d'agriculture paysanne favorisant une alimentation locale, respectueuse de la nature et soucieuse du bien-être de l'animal, mais aussi des acteurs du monde paysan, il apparaît nécessaire d'accompagner ces derniers dans la transition vers un élevage et un abattage éthiques. À cet égard, il convient particulièrement d'accompagner ceux qui dépendent aujourd'hui de l'élevage intensif, afin de leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Selon un sondage réalisé par l'IFOP en janvier 2021, quelque 85 % des Français se déclarent opposés à l'élevage intensif, signe que l'opinion publique est favorable à la mise en place de cette nécessaire transition. Cette évolution de l'opinion, nous la devons aussi au travail des lanceurs d'alerte et aux actions des associations. Au niveau européen, la directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages pose les grands principes du bien-être chez les animaux domestiques de production pour les États membres s'agissant des bâtiments et infrastructures, de la liberté de mouvement, de l'alimentation, des mutilations et maltraitances. Elle n'en détaille cependant pas la mise en oeuvre et laisse aux États membres une large marge d'action.

les taux respectifs de 83 % et 69 %. La France, elle, n'arrive qu'en dix-septième position de ce classement, avec un score de 25 %, derrière la Roumanie, la Croatie et la Hongrie. Nous devons instaurer en Europe un étiquetage alimentaire transparent, comprenant un descriptif clair du mode d'élevage, de sorte que le consommateur-citoyen puisse pleinement jouer son rôle dans la protection du bien-être animal, ainsi que de sa santé et de l'environnement, sans, bien sûr, léser économiquement les agriculteurs, qui doivent pouvoir résister aux importations issues de pays qui ne suivent pas le même cahier de charges en termes de conditions sanitaires, de bien-être animal et de respect de l'environnement, par exemple en instituant Les agriculteurs sont les premiers à pâtir de l'élevage industriel, déjà au niveau économique, avec la réduction du nombre d'exploitations et la concentration d'élevages toujours plus importants Quant aux niveaux éthique et moral, je le rappelle, les agriculteurs aiment leurs bêtes et voudraient s'assurer de leur donner, autant que possible, « une bonne mort », sans souffrance. de loi, étant donné la relative brièveté du temps de débat qui lui est imparti, n'aborde pas en détail la question de l'abattage, tout en soulignant les vertus possibles de l'abattage de proximité. Son article 1 tend à garantir progressivement, d'ici à 2040, un accès extérieur et une surface par tête adaptés, en tenant compte des moments de vie de l'animal et des cas spécifiques, géographiques ou climatiques, comme les élevages en montagne, à l'horizon de 2040, avec une mise en place progressive des dispositifs d'accès au plein air et des seuils de densité maximale dès 2025. L'article 2 limite la durée de transport des animaux à huit heures sur le territoire national, dans des conditions assurant leur bien-être. L'article 3 interdit l'élimination, sauf en cas d'épizootie, des poussins mâles et des canetons femelles vivants. Broyés, étouffés, gazés, les poussins mâles sont victimes d'un cauchemar industriel, lequel est, hélas, toujours une réalité en France. L'Allemagne confirme sa position de pionnière dans la lutte contre le broyage et le gazage des poussins mâles en interdisant cette pratique Un projet de loi a été validé vendredi dernier par le Bundestag. Le sexage sera pratiqué en amont, entre le neuvième et le quatorzième jour, pour déterminer le sexe des embryons.

faut-il que cette promesse soit tenue ! La filière des oeufs annonce qu'elle ne sera pas prête pour cette date, mais se prépare timidement à se lancer dans le déploiement du sexage. Nous demandons, quant à nous, l'interdiction de l'élimination Le passage à l'élevage éthique nécessite l'accompagnement financier des agriculteurs. Pour cette raison, notre texte prévoit un fonds pour les aider à transformer leur activité et à se conformer au nouveau cadre juridique, y compris en développant l'abattage de proximité. La puissance publique a un rôle crucial à jouer dans la transition écologique. Subventionner les investissements des agriculteurs par des prêts à taux zéro ou garantis par l'État figure parmi les quelques solutions envisageables. Notre pays vit une urgence sociale, sanitaire, climatique et environnementale. Il vit aussi dans une urgence éthique. Nos jeunes, défilant nombreux dans nos rues pour le climat, ne cessent de nous le rappeler. Il est donc primordial, mes chers collègues, d'engager sans délai cette démarche vers un modèle respectueux du vivant. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat, nous permettant d'avoir un débat de société sur le thème du bien-être animal. Je crois que tous les parlementaires ici- je dis bien « tous » -partagent vos préoccupations. Les bonnes pratiques en matière d'élevage, de transport et d'abattage sont un souci de tous les jours, qui prendra une place de plus en plus importante dans les années à venir. La société et les filières le veulent, et c'est bien normal. Tous les parlementaires, comme toutes les filières, veulent tendre vers plus d'élevages alternatifs à la cage ou au bâtiment. Nous voulons tous améliorer les conditions de transport des animaux : c'est un sujet consensuel, ce que montre d'ailleurs l'adoption très large et transpartisane de résolutions du Parlement européen sur le sujet. Enfin, il faut bien entendu trouver une solution viable au broyage massif de poussins. C'est justement la raison pour laquelle la commission partage pleinement vos objectifs, mais en contestant fermement les moyens retenus et, surtout, les effets de bord importants induits par la rédaction de la proposition de loi.

pour perdre de l'argent, personne ne peut le supporter. C'est ce qui explique que la décapitalisation du cheptel se poursuive dans certaines filières. Si la situation perdure, notre souveraineté alimentaire en élevage est menacée, d'autant que les importations sont déjà très présentes 45 % de notre consommation de poulet, 25 % pour le porc, 55 % pour les ovins et un tiers de nos produits laitiers. Si rien n'est fait, nous perdrons les externalités positives de notre élevage en matière d'aménagement du territoire, de stockage de carbone, de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels de biodiversité des races cultivées ... Ce contexte devait être rappelé pour garder à l'esprit qu'il faut être à l'écoute de nos éleveurs. Lors de nos auditions,

Des élevages expérimentaux se développent pour éviter l'élevage de lapins en cage. Rappelons aussi que 94 % des vaches laitières et 67 % des vaches allaitantes ont accès à l'extérieur. La France est

et développent des outils de diagnostic sur les exploitations, afin de mieux mesurer les progrès à réaliser. Cette situation doit être dans tous nos esprits à l'heure d'examiner des propositions pour interdire certaines pratiques d'élevage, de transport ou d'abattage. Ces rappels étaient d'autant plus nécessaires que l'intitulé de la proposition de loi ignore cette réalité : en plaidant « pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal », il est sous-entendu qu'il n'existe pas d'élevage éthique et soucieux du bien-être animal aujourd'hui en France. Je veux le dire clairement : cela ne correspond pas à la réalité du terrain agricole. La proposition de loi pose également des difficultés pratiques. En ce qui concerne l'élevage en plein air, par exemple, l'article 1 entend interdire toute construction de nouveaux bâtiments d'élevage ne prévoyant pas un accès à l'extérieur des animaux à compter de 2026 et interdire tout élevage et interdire tout élevage qui ne soit pas en plein air à horizon de 2040. Soit ! Mais les instituts techniques des filières rappellent que cette généralisation pose des difficultés en matière de bien-être animal pour certaines espèces, ainsi que des interrogations en matière de biosécurité. On l'a vu récemment avec l'influenza aviaire : le tout plein air expose à davantage de risques épidémiques. Notre résilience et notre souveraineté se jouent dans la complémentarité de nos élevages, non dans leur opposition. J'ajoute que le plein air impliquerait la mise en place d'un parcours pour les animaux qui est fortement consommateur de foncier. Rien que pour le porc, le passage au tout plein air en 2040 représente une consommation foncière équivalente à un département français. Pour les poules pondeuses, il faudrait trouver l'équivalent de la surface de la ville de Paris. Quand on connaît les difficultés liées à l'artificialisation des sols, je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes

J'ajoute que la proposition d'article 2, conformément au droit européen, ne réglemente les durées de transport que sur le territoire national. Dès lors, si un camion traverse une frontière, la réglementation française ne lui sera plus applicable applicable et il bénéficiera d'une réglementation européenne moins-disante. Il sera donc pertinent économiquement pour lui de s'approvisionner auprès d'abattoirs étrangers, faisant faire plus de route aux animaux. Il me semble que c'est le contraire de l'objectif de la loi De même, les bassins de production sont parfois très éloignés des abattoirs ou des couvoirs. En limitant, par exemple, la durée des transports à quatre heures pour la volaille et le lapin, dont les abattoirs et les couvoirs sont presque exclusivement à l'ouest de notre pays, on s'interdirait tout élevage ailleurs que dans que dans cette région en France : est-ce ainsi que nous favoriserons les circuits courts et la diversification de notre agriculture ? De plus, la commission des affaires économiques a estimé que l'échelle d'action n'était pas la bonne, car la question doit, dans son ensemble, être portée au niveau européen. À défaut, on alourdirait encore les contraintes sur nos agriculteurs français, tout en exportant les pratiques que la loi condamnera chez nos voisins, ce qui se traduirait par davantage d'importations de denrées. Cela ne ferait aucun gagnant en matière de bien-être animal, réduirait notre souveraineté alimentaire et dégraderait le bilan environnemental de notre alimentation. J'en veux pour preuve la délicate question du broyage et du gazage des poussins mâles et des canetons femelles. Les techniques de recherche de sexage dans l'oeuf ont considérablement évolué et permettent effectivement d'envisager de tourner la page du broyage à court terme. Oui, il faut s'en féliciter, mais imposer une interdiction intégrale dans huit mois, c'est condamner des petits couvoirs et c'est surtout renchérir le coût des ovoproduits issus d'élevages français, qui représentent 40 % de la production totale. Or, pour ces produits, l'aspect prix est essentiel : à aller trop loin, nous renforcerions la compétitivité des ovoproduits polonais, qui inonderaient notre marché, alors que les poussins continueraient, en Pologne, à être broyés. Pour le broyage des poussins, je crois qu'il faut faire confiance aux accouveurs. Le marché est prêt, la recherche évolue et se perfectionne. Je suis sûre que nous y parviendrons dans un laps de temps bref. Les filières ont d'ailleurs renouvelé leurs engagements sur l'oeuf coquille à très court terme. Faisons-leur confiance. L'Union européenne doit nous faire évoluer collectivement pour limiter les distorsions de concurrence et pour que ces mesures soient réellement efficaces. Monsieur le ministre, je vous interroge : quels engagements le Gouvernement

Enfin, j'entends, bien sûr, les critiques de certains qui trouvent, au contraire, que la loi est équilibrée, dans la mesure où elle prévoit une compensation par un fonds pour les pertes induites par la présente proposition de loi.

d'interdiction sans aide. Toutefois, l'analyse a démontré que la création de ce fonds était irréaliste, car les chiffres des surcoûts induits par la proposition de loi sont colossaux : rien que pour le porc, le surcoût du plein air est estimé à 13 milliards d'euros.

de la PAC, une échéance majeure pour tous nos agriculteurs. Chacun sait ici que le bien-être animal et le respect de l'environnement sont des sujets essentiels pour nos concitoyens. Sur ces questions, les débats pointent trop souvent du doigt les éleveurs français, alors qu'ils sont les premiers à souhaiter plus de bien-être animal. En faisant le pari de la modernisation des infrastructures d'élevage et d'abattage, le Gouvernement agit avec méthode et pragmatisme, aux côtés de nos éleveurs, pour leur donner les moyens de répondre aux attentes sociétales. Ces sujets de long terme nécessitent une politique d'accompagnement, et non des bouleversements radicaux.

le seul prisme de l'émotion. Madame la sénatrice Esther Benbassa, soyez en assurée, le Gouvernement partage votre ambition d'améliorer les conditions d'élevage, de transport ou d'abattage au sein de la grande ferme France. ferme France. Il aborde ces enjeux de transition avec raison et pragmatisme. Nous devons répondre aux impératifs biologiques des espèces et définir collectivement les modalités les plus adaptées pour répondre au bien-être des animaux,

En premier lieu, je souhaite rappeler que les élevages français sont à taille humaine, bien loin des élevages industriels qui existent ailleurs dans le monde. Ensuite, l'élevage français est l'un des plus durables au monde. Les filières mettent tout en oeuvre pour assurer la transition agroécologique. Les plans de filière mis en place à partir de 2017 ont déjà prouvé leur efficacité. Sur le plan sanitaire, prenons l'exemple de la lutte contre l'antibiorésistance le plan porté par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a porté ses fruits, avec une réduction de 37 % des utilisations d'antibiotiques en cinq ans. L'exposition des animaux aux antibiotiques, en France, est inférieure à la moyenne européenne. Assurer un minimum d'accès au plein air à tous les animaux d'élevage dès 2040 n'est pas raisonnable. Prenons quelques exemples factuels. Le plein air représente aujourd'hui 5 % de la production. Aujourd'hui, ce sont 82 % de la production de poulets de chair qu'il faudrait repenser.

laisser croire que, dans vingt ans, nous n'aurons plus aucun poulet ni porc standard dans nos fermes est faux et contreproductif si cette ambition n'est pas réfléchie à l'échelle du marché unique et des relations commerciales internationales. Le temps de l'agriculture est long. Il faut assurer des transitions adaptées au marché, sans quoi nous serons rapidement confrontés à une augmentation de produits importés à moindre coût venant de pays qui ne respectent pas nos pratiques, notamment de viandes provenant d'élevages très intensifs. Le débat sur le transport des animaux vivants doit également s'inscrire dans cette réflexion, laquelle doit avoir lieu à l'échelle au moins européenne, pour éviter tout effet de concurrence déloyale au détriment des opérateurs qui travaillent exclusivement sur le territoire national.

dans le courant de 2021, sans qu'une modification législative soit nécessaire. J'ajoute que le plan de relance et son volet relatif à la modernisation des abattoirs favoriseront aussi des filières locales et auront donc un effet indirect bénéfique sur le transport des animaux vivants. qui concerne les transitions et l'amélioration du bien-être animal, la fin du broyage des poussins est un exemple concret des enjeux auxquels nous devons répondre. La filière oeufs et les couvoirs, principaux impactés par cette transition, bien intégré l'objectif et l'attente des citoyens en la matière. La question de la formalisation de l'interdiction est finalement secondaire aujourd'hui, car des méthodes opérationnelles existent. L'enjeu est de savoir qui paie le coût de cette transition. L'État, au travers du plan de relance, peut engager des changements en finançant une partie des investissements, mais un modèle pérenne ne peut pas reposer exclusivement sur lui. Le coût de la transition implique également des changements de pratiques au quotidien. La filière travaille sur une feuille de route opérationnelle. En outre, inscrire une mesure d'interdiction dans la loi ne permettrait pas d'accompagner financièrement les filières,

que, au cours des dernières années, nous avons imposé énormément de nouvelles contraintes aux éleveurs français pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Restons sur l'exemple criant de la filière poules pondeuses

C'est tout le sens de notre action. Les États généraux de l'alimentation ont permis d'améliorer la structuration des filières, avec des exigences accrues en termes de respect de l'environnement et du bien-être animal, reposant sur des signes de qualité. Je tiens ici à saluer la responsabilisation des professionnels, qui se sont organisés autour de plans de filière et de chartes de bonnes pratiques, pour répondre aux attentes sociétales. Une véritable transition est en marche. Toute transition a un coût et nécessite un accompagnement réfléchi. Le plan France Relance consacre ainsi près de 300 millions d'euros à la modernisation de nos élevages et de nos abattoirs et à la structuration des filières, afin d'accélérer cette transformation. cette montée en gamme ne peut pas uniquement reposer sur la responsabilisation des professionnels et l'accompagnement du Gouvernement. Les injonctions des citoyens doivent se traduire dans leurs actes d'achats. C'est tout le sens de la loi Égalim, dont l'objectif est d'aboutir à une meilleure rémunération des agriculteurs. Nous devons sortir de la guerre des prix bas. Il n'est pas possible de demander toujours plus aux éleveurs sans leur en donner les moyens.

seulement en accompagnant nos éleveurs que ces derniers pourront créer de la valeur et faire face aux grands enjeux de société. Comme toute transition, celle-ci n'aura pas lieu sans un changement profond des mentalités, c'est-à-dire tant que les éleveurs seront forcés de produire toujours moins cher.

messieurs les sénateurs : même si l'agenda du Sénat est particulièrement chargé- vous le savez mieux que moi -, je vous confirme l'intention du Gouvernement de voir ce texte inscrit à l'ordre du jour de vos travaux avant la fin de l'année. Le Gouvernement est mobilisé et souhaite préserver notre modèle d'élevage équilibré, qui se distingue par des exigences parmi les plus fortes au monde. Mais là où certains mènent une campagne de dénonciation et de stigmatisation généralisant trop souvent des cas isolés, nous revendiquons une politique de mesures concrètes, en agissant sans trembler quand cela s'impose, mais sans jamais jeter injustement l'opprobre sur tout un secteur ou toute une filière. le Gouvernement tient à saluer le travail mené par Henri Cabanel et Françoise Férat sur l'accompagnement de la détresse, longtemps ignorée, Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons rejeter la radicalité qui mettrait fin à l'élevage français par excès d'exigence. Je le répète, nous partageons la volonté de poursuivre l'amélioration des bonnes pratiques, mais je vous invite à faire preuve de raison et de bon sens. La question de l'avenir de l'élevage suppose beaucoup d'ambition et de pragmatisme, mais aussi et surtout de confiance en nos éleveurs, qui sont indiscutablement les premiers à souhaiter agir pour le bien-être des animaux et pour l'environnement. Ils travaillent chaque jour pour nous fournir la meilleure alimentation possible. Ce n'est pas en les stigmatisant que nous aboutirons à un élevage plus durable, mais en leur donnant les clés pour mener des transitions ambitieuses. seulement en mettant la question de la rémunération des éleveurs au centre des discussions que nous pourrons accélérer le changement durable que nous appelons de tous nos voeux. Refuser cet état de fait, c'est condamner nos éleveurs.

une proposition de loi peut-elle, en quelques bonnes intentions, changer le monde ? C'est la question que je me pose souvent lors de l'examen de textes touchant à des enjeux sociétaux. Ce débat qui nous réunit aujourd'hui en fait partie comment être contre des objectifs d'élevage éthique, rémunérateur, socialement juste et soucieux du bien-être animal ? Comment être contre l'interdiction de l'élimination de poussins mâles et de canetons femelles vivants ? Je remercie le groupe Écologiste - Solidarité et territoires de porter au débat des objectifs aussi nobles. Cependant, je m'interroge sur l'opportunité de ce texte, alors que le mal-être des agriculteurs n'a jamais atteint un tel paroxysme : deux agriculteurs se suicident chaque jour ; ne les oublions pas. Si vous l'évoquez dans l'exposé des motifs en pointant un élevage intensif, qui ne respecte ni les agriculteurs ni les animaux, les mettant ainsi au même niveau, je souhaite poser ici un préambule

Notre société ne parvient plus aujourd'hui- plus encore avec les réseaux sociaux, qui réduisent les débats à néant, qui sclérosent la pensée, qui la congestionnent en un « pour ou contre » -à comprendre les enjeux et les conséquences de décisions parfois irrémédiables.

Cette posture ne mènera à rien, sinon à l'ascension des extrêmes. C'est la raison pour laquelle il faut appréhender les problèmes de façon globale, réunir toutes les parties prenantes et agir avec l'ensemble des postulats, loin des passions et des fantasmes. J'aime répéter que l'agriculture, ce n'est pas un enjeu, mais un faisceau d'enjeux- environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux, mais aussi de santé publique, d'indépendance alimentaire ... -, qu'il faut traiter de façon transversale. Privilégier un axe plutôt qu'un autre déséquilibre nos filières déjà bien fragilisées par les crises sanitaires, climatiques et économiques successives, ainsi que par une perte de compétitivité due à une surtransposition des règles européennes. Je m'inquiète réellement des effets des lois qui n'ont de conséquences que sur les paysans français. J'estime que les enjeux légitimes que vous posez doivent être examinés et votés au niveau européen. limiter les mesures aux éleveurs français équivaut à instaurer, de fait, une concurrence déloyale entre les filières des États membres. Toute interdiction de mode de production va isoler nos agriculteurs dans un marché européen déjà très concurrentiel et,, au sein d'un marché mondial libéral, où le prix le plus bas s'oppose aux modes de production durables. Vous le savez, je prône les circuits courts et les signes de qualité. Mais, alors que nos agriculteurs travaillent en moyenne 55 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1 036 euros, soit 4,7 euros de l'heure, je pense qu'il faut nous poser avant de trancher dans le vif. d'agriculteurs s'est d'ailleurs déjà tourné vers des pratiques vertueuses. Avez-vous analysé l'impact de votre texte sur la compétitivité des filières ? Avez-vous analysé l'impact financier des mesures d'accompagnement ? Avez-vous réellement analysé l'impact sur le bien-être animal ? En effet, les consommateurs qui mangent de la viande à bas prix se tourneront vers des produits étrangers. Nous n'aurons alors aucune possibilité de connaître les conditions de vie et d'abattage des animaux, ce qui réduira quasiment à néant Je suis sincèrement persuadé que c'est non pas une loi, mais bien une évolution des mentalités qui changera le monde. Associer le consommateur à l'acte d'achat, lui faire prendre conscience que son choix n'est pas anodin et qu'il peut agir sur les modes de production : tout cela est fondamental. Aucune loi ne pourra remplacer ce libre arbitre. Il faut donc accompagner le consommateur. L'étiquetage lui fournit les informations dont il a besoin. Les applications, les QR codes, le Nutriscore se développent, et la filière agroalimentaire répond à la poussée sociétale à laquelle les agriculteurs s'adaptent déjà.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question du bien-être animal comporte des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, culturelles, sociales, religieuses et politiques. Elle transcende tous les courants de pensée. Nos Nos concitoyens et concitoyennes y sont de plus en plus sensibles. Nous ne pouvons nier les alertes lancées sur la violence des conditions d'élevage, de transport et d'abattage dans certains endroits, même si certains ne voudraient pas le voir, quand d'autres voudraient le cacher. La maltraitance dans certains abattoirs, ... Certains ! ... l'élevage en batterie et le broyage des poussins interrogent notre modèle agro-industriel, mais aussi, plus largement, notre modèle de société. ce que nous infligeons aux animaux est un miroir sombre, sur lequel il ne fait pas bon se pencher. La pression productiviste et les inégalités s'intensifient pour les humains comme pour les animaux. Songeons à la violence subie par les animaux d'élevage intensif. Mais songeons aussi à la violence subie par le personnel des abattoirs ou à celle des licenciements massifs par des groupes peu scrupuleux lancés dans la course au profit. Je pourrais égrener de nombreux exemples. Accepter la possibilité de maltraiter, quel que soit l'être maltraité, c'est ouvrir une brèche vouée à se creuser ; c'est créer un précédent dans la violence et l'aliénation ; c'est vouloir détruire l'altérité. L'alimentation est à la fois une nécessité vitale, un plaisir et un moment de convivialité avec nos proches. Mais à l'heure de la crise environnementale et de l'industrialisation de l'élevage, nous n'avons d'autre choix que d'intégrer aussi sa dimension éthique. Repenser le rapport de l'humain à la nature et au monde animal, est une nécessité. Toutefois, nous pensons qu'il faut sortir de la vision binaire « pour ou contre » l'élevage ou la viande, pour poser la question du modèle d'élevage et d'agriculture que nous voulons. L'émergence de la question du bien-être animal frappe un secteur déjà fragilisé par les crises sanitaires et économiques de ces dernières décennies. Mais défendre l'élevage, c'est reconnaître les dérives entraînées par le modèle hyperproductiviste, soit 80 % de l'élevage en France, qui nuit à l'ensemble des éleveurs. En 2019, le Conseil économique, social et environnemental alertait sur ces transformations et sur la baisse de rémunération qui les accompagne. Ainsi, en trente ans, le nombre d'éleveurs a chuté de 57 % dans le secteur des porcs et volailles et de 70 % dans celui des vaches laitières. Cet effondrement n'a pas empêché les cheptels d'augmenter, ni les animaux d'être abattus en masse. C'est l'agriculture paysanne qui est la première victime, au profit de fermes des « mille vaches ». France Nature Environnement pointe la concentration croissante, qui entraîne des risques sanitaires, et l'impact environnemental. La multiplication des accords de libre-échange, pression supplémentaire pour nos agriculteurs, et sur eux, exacerbera encore ce phénomène.

et la recherche de meilleures conditions d'élevage. La plupart des réglementations et cahiers des charges nationaux et européens visant à protéger les animaux sont basés sur les cinq libertés du rapport Brambell, qui date déjà de 1965. Il s'agit d'assurer l'absence de faim et de soif, d'inconfort, de douleur, de blessures et de maladie, de peur et de détresse, ainsi que de garantir un espace suffisant et adapté et la compagnie d'autres congénères. principes ne sont pas contraignants et les moyens manquent pour assurer les contrôles et permettre à nos éleveurs de réaliser cette transition. C'est tout l'intérêt de l'article 4, qui propose un fonds dédié à cette transition, dans une vision longue. Il faut aller plus loin et passer d'un élevage intensif, industriel et destructeur, à un élevage respectueux de l'environnement, de l'humain et de la planète.

le développement de nombreuses associations de défense des animaux et les actions « coup de poing » qu'elles ont pu mener ces dernières années sont des manifestations de l'importance que revêt le bien-être des animaux dans l'opinion publique. Nous avons vu les images choquantes de certains abattoirs, diffusées sur les réseaux sociaux, et nous n'y sommes pas insensibles, mais permettez-moi également de penser aux hommes qui y travaillent. Le constat posé par cette proposition de loi met en lumière de véritables enjeux sociétaux, que nous ne devons pas négliger. Rappelons que les éleveurs, dans leur très grande majorité, réprouvent ces traitements ignobles. Ils respectent au quotidien le bien-être de leurs animaux, que les exploitations soient petites ou grandes. Ils appliquent scrupuleusement les normes européennes et nationales, pour assurer de bonnes conditions à leurs bêtes. Ils ont investi des centaines de milliers d'euros pour adapter leurs étables et leurs porcheries- jusqu'à la prochaine norme Soyons clairs : s'ils sont avérés, les manquements au bien-être animal doivent être sanctionnés. Les intentions de ce texte sont louables, et l'Union Centriste partage la volonté d'améliorer les conditions de travail des éleveurs et le bien-être des animaux de ferme. Malheureusement, les solutions avancées dans cette proposition de loi ne répondent pas aux problématiques profondes de la filière. Ce texte risque de mettre un peu plus à genoux financièrement nos producteurs qui respectent les règles.

D'un point de vue technique, le tout plein air n'est pas faisable : l'accès au foncier sera un facteur limitant pour nombre d'éleveurs. Ces mesures vont fragiliser les filières, et les agriculteurs qui ne parviendront pas à réaliser les investissements nécessaires cesseront leur activité, sans repreneur. Il ne faut pas que la généralisation du plein air en fasse le nouveau standard, au détriment de la rémunération du producteur. Sans consentement du consommateur à payer le coût du changement de pratiques, cette mesure encouragera les importations.

De plus, si nous rendons l'élevage en plein air systématique, nous faciliterons la diffusion d'épidémies animales. Quelles dispositions seront prises pour contrer la propagation éventuelle de la peste porcine ? Comment empêcher les contacts avec la faune sauvage, vecteur de grippe aviaire ? de même des modifications proposées pour les transports d'animaux à l'article 2 : si nous limitons à quatre heures les transports dans l'Hexagone, comment s'assurer que les camions ne feront pas de détours par l'étranger ? Quelle sera la facture carbone de telles dérives ? Sur le papier, tout est très simple ; mais sur le terrain, ces solutions ne sont pas fonctionnelles. L'enjeu prioritaire pour assurer le temps de transport le plus réduit possible est de renforcer un maillage d'abattoirs de proximité économiquement viables et sanitairement fiables. le dispositif proposé n'est pas viable financièrement. Dans la filière porcine, la construction de bâtiments offrant un accès au plein air- courettes, différent d'élevage plein air -coûterait 13 milliards d'euros pour l'ensemble du cheptel. Le budget nécessaire pour accompagner la transition par rapport aux moyens disponibles rend ces mesures irréalistes. À titre de comparaison, le plan de relance prévoit une enveloppe de 100 millions d'euros pour l'ensemble de la mesure « Biosécurité et bien-être animal ». Tout cela est bien insuffisant pour une telle transition. La France devra-t-elle créer une nouvelle taxe et pénaliser la compétitivité de notre filière nationale ? Ce dispositif n'est pas viable non plus pour les éleveurs. N'oublions pas en effet que ces restructurations ont un prix et que tous les producteurs ne seront pas éligibles aux aides du fonds de soutien. derniers, ce sera la double peine : ils devront s'endetter pour financer des investissements qu'ils n'amortiront pas à court terme et augmenter le prix de leurs produits, déjà peu compétitifs sur le marché international. Sachant qu'un Français sur sept saute des repas pour des raisons financières, vous comprendrez aisément que le consommateur moyen pourrait encore plus facilement porter son choix vers le porc espagnol, deux fois moins cher que le porc français.

La France a présenté un travail commun avec l'Allemagne pour parvenir à une solution viable pour la filière d'ici à la fin de 2021, date d'interdiction de cette pratique. Enfin, chers collègues, n'oublions pas les efforts déjà consentis en matière environnementale et sociétale par l'agriculture en général et l'élevage en particulier, efforts trop souvent oubliés au profit d'un agribashing grandissant et agressif. Je témoigne ici, au nom du groupe Union Centriste, que la ferme France est la meilleure du monde. Contraindre une fois de plus l'élevage français aggravera la situation de détresse à laquelle certains sont confrontés.

Travaillons pour convaincre nos compatriotes qu'une viande de qualité, respectant le bien-être animal, requiert un prix d'achat décent.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le néolithique, qui vit la sédentarisation se développer et l'élevage apparaître dans de nombreuses régions du monde, l'homme a évolué dans une relation à la fois constructive et problématique avec l'animal, que ce dernier soit mythique, sauvage ou élevé à des fins nourricières ou d'auxiliaire de travail. Portée par la pensée, de l'Antiquité à nos jours, la nature de cette relation a été interrogée dans le cadre de la religion, de l'éthique et de la morale, de l'économie et du droit en général, de la nature et des droits particuliers que nous lui avons progressivement reconnus. Je ne rappellerai pas les grandes étapes de ce cheminement intellectuel, mais on sait qu'il était déjà présent dans l'Antiquité, que d'aucuns considèrent, chimériquement peut-être, comme l'âge d'or de la relation entre l'homme et l'animal. De ce long cheminement, qui a connu des inflexions importantes en Angleterre, au XVII siècle, et en France au moment des Lumières, avec Condillac et son prémonitoire, deux concepts différents ont émergé : celui du « droit de l'animal » et celui du « bien-être animal

Mais y souscrire ne laisse pas entendre que rien n'est fait aujourd'hui en ce sens ou que les éleveurs et industriels français ne s'en soucient pas. Comme beaucoup ici,

Ils sont attendus par une grande partie de la société et ils le savent. Comme le montrent les études, le sujet est sociétal et prend de plus en plus d'importance dans les consciences des citoyens et des consommateurs.

Dans le cadre juridique actuel, il faut se donner les moyens de contrôler et de sanctionner comme il se doit les fautifs. Monsieur le ministre, c'est votre rôle et votre responsabilité. De la même De la même manière, nous nous interrogeons sur les suites données aux « mesures pour la protection et l'amélioration du bien-être animal », proposées aux interprofessions par le Gouvernement en janvier 2020.

renforcer la sensibilisation et la formation au bien-être animal ; améliorer la qualité de vie des animaux d'élevage ; améliorer les conditions de transport des animaux ; améliorer l'information des consommateurs ; responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie. Monsieur

l'article 1,demandant au Gouvernement de remettre au Parlement un bilan, un état des lieux exhaustif de l'ensemble des démarches engagées en faveur du bien-être animal en France, pour évaluer leur efficacité. Ce bilan informera sur les actions mises en oeuvre dans le monde de l'élevage, mais aussi sur celles qui sont portées par la société civile ou les entreprises. panorama précis permettra aux pouvoirs publics, mais également à l'ensemble des acteurs mobilisés sur cette question, de savoir réellement où la France se situe en matière de bien-être animal et de déterminer les mesures proportionnées à mettre en oeuvre pour accompagner et, si nécessaire, accélérer ce mouvement. Pour avoir un débat apaisé sur la question du bien-être animal, nous devons savoir précisément d'où nous partons, réellement et objectivement, pour mettre en oeuvre des actions ou des politiques ciblées et efficaces. Enfin, nous tenons à rappeler notre attachement à l'élevage, à ce qu'il représente pour nos territoires- je viens moi-même du Gers, une zone de polyculture et d'élevage qui souffre beaucoup

... Parce qu'ils sont en première ligne de la souffrance, nous proposerons, à l'article 4, que les aides prévues servent également à la mise en oeuvre de mesures de soutien et d'accompagnement psychologique pour les agriculteurs, sans oublier les opérateurs de l'abattage, afin de leur apporter une écoute et de leur proposer des mesures améliorant leur « bien-être au travail » et leur bien-être tout court d'hommes et de femmes, de travailleurs dignes de respect et de considération.

je tiens à saluer le travail mené par notre collègue Esther Benbassa, en lien avec Mme la rapporteure de la commission des affaires économiques, Marie-Christine Chauvin. Elles ont réalisé un travail complet, en consultant les acteurs des filières. Cette proposition de loi permet d'ouvrir un débat important, en discutant d'options concrètes et pas seulement d'idées abstraites. Je le dis au nom du groupe Les Indépendants - République et Territoires : nous partageons les préoccupations de notre collègue pour valoriser le travail

Avant d'exposer les raisons de notre désaccord sur ce texte, je tiens à saluer les efforts continus de nos agriculteurs pour adapter leurs méthodes de travail aux nouvelles préoccupations et attentes sociétales et environnementales. Toutes ces évolutions vont dans le bon sens. À cet égard, la France s'inscrit dans une dynamique européenne partout sur le continent nos agriculteurs s'adaptent, pour mieux prendre en compte les attentes des consommateurs en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement et de bien-être animal. L'agriculture française, il faut le dire et le marteler, est l'une des plus durables au monde. Sur bien des aspects, nous sommes en avance. Nous pouvons en être fiers, mais nous aurions tort de réfléchir dans un cadre franco-français : notre agriculture doit aussi veiller à rester compétitive, en évitant de faire émerger des distorsions de concurrence, notamment entre pays européens. C'est C'est en conquérant des marchés à l'international et en réalisant des investissements productifs que notre agriculture pourra conserver son excellence, sa robustesse, et contribuer pleinement à la souveraineté et à la sécurité alimentaires de la France.

Lors du dernier budget, nous étions nombreux à soutenir la modernisation des abattoirs et des élevages dans le cadre du plan de relance. Cela montre que nous pouvons améliorer notre performance économique en intégrant le bien-être animal. En conclusion, je rappellerai que nous devons aussi nous préoccuper du bien-être des éleveurs, qui aiment leurs animaux. Leur métier est difficile et exigeant

C'est aussi un enjeu pour les agriculteurs, qui vivent au quotidien avec leurs animaux. Nombre d'éleveurs peinent aujourd'hui à trouver un équilibre économique et se retrouvent face à une société qui leur demande des changements coûteux en termes d'investissement et de temps pour réorienter leur pratique. Toutefois, il y a pire : les éleveurs dits « intégrés », qui n'ont pas le choix.

Alors, il nous faut agir collectivement, pour donner aux éleveurs les moyens de la transition. Pour ce faire, nous devons fixer un cap clair : c'est ce que nous proposons dans cette proposition de loi, avec pour objectif un élevage donnant accès au plein air

qui serait gagnant si nous substituions aux produits issus d'élevages industriels français des produits issus d'élevages bien plus intensifs, mais situés ailleurs et ne respectant pas nos normes ?

les projets alimentaires territoriaux et par la création de débouchés rémunérateurs, la restauration collective. Malheureusement, aujourd'hui encore, le plan de relance est loin d'être suffisant dans ce domaine. Il faut enfin, en parallèle, travailler à l'accessibilité pour toutes et tous de produits qui sont plus respectueux des animaux et de l'environnement, mais aussi plus rémunérateurs pour les éleveurs. Là encore, nous pouvons et nous devons nous donner les moyens d'y parvenir, en rémunérant en rémunérant les externalités positives générées par les élevages respectueux du bien-être animal et de l'environnement et en travaillant sur le droit à l'alimentation pour tous, en particulier sur la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Il nous faut tout mettre en oeuvre en oeuvre, aujourd'hui, pour réussir en urgence une transition vers un élevage éthique et respectueux des éleveurs, des animaux et de l'environnement. On parle beaucoup de fractures dans notre pays ; on en connaît plusieurs. dans le monde agricole aussi, une fracture est en train de se creuser, entre ceux qui souhaitent la poursuite de l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage et ceux qui pratiquent et défendent une agriculture paysanne, génératrice d'emploi, de développement local et de respect du climat, de la biodiversité, des animaux et des êtres humains.

sait, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions ! Tout d'abord, le choix du titre de votre proposition de loi n'est pas anodin. Il favorise le soupçon à l'égard des agriculteurs, ce qui est regrettable. qu'agricultrice, je puis vous assurer que la très grande majorité des membres de notre profession placent le bien-être de leurs animaux au coeur de leurs préoccupations.

l'interdiction, au 1 janvier 2026, de la construction ou de l'extension de bâtiments d'élevage si la densité de peuplement n'est pas limitée et que l'accès à un espace de plein air n'est

l'interdiction de l'élimination, sauf en cas d'épizootie, des poussins mâles et des canetons femelles vivants, à partir de 2022. Ces interdictions et limitations font fi des efforts réalisés et fixés par les différentes filières pour améliorer le bien-être animal. Elles se limitent au cadre national, alors que l'échelle idoine est européenne.

ces interdictions et limitations, on fait comme si le Gouvernement n'avait pris aucune mesure concrète pour améliorer le bien-être des animaux d'élevage. Au contraire, la mobilisation gouvernementale a permis d'acter, sans légiférer, l'interdiction de la castration à vif des porcelets et de l'élimination à terme des poussins mâles dans la filière pondeuse. l'article 4 de cette proposition de loi, qui crée un fonds de soutien pour le bien-être animal, il est déjà satisfait : le plan de relance permet à l'État d'apporter des financements pour accélérer la transition vers un modèle agricole respectueux du bien-être animal.

Cela se traduira concrètement par la création d'une bergerie avec des mangeoires et des abreuvoirs, la mise en place de quais d'accessibilité, l'extension de l'abattoir pour améliorer le confort des animaux, l'installation d'un système de vidéosurveillance et la mise en place de formations sur le bien-être animal pour les salariés. Pour toutes ces raisons, en responsabilité, notre groupe ne pourra pas voter en faveur de ce texte. Pour ma part, comme un certain nombre de mes collègues, je m'y opposerai.

Bien sûr, il y a des sujets sur lesquels nous pouvons ouvrir le débat. Joël Labbé a bien dit- je l'en remercie -qu'il y a peut-être des questions à se poser

une agriculture familiale. C'est cela qu'il faut continuer de défendre, c'est cela qu'il faut continuer de préserver. Or ce n'est pas en condamnant cette

En fait, nous n'en avons pas débattu depuis l'examen nocturne de quelques articles de la loi Égalim, qui contenaient des dispositions sur les poules pondeuses et une expérimentation de captation vidéo dans les abattoirs. Il en était évoqué une dizaine, sur la base du volontariat ; il y en aurait aujourd'hui quatre tout au plus, ce qui montre d'ailleurs tout l'allant du Gouvernement sur ces questions. Il faut donc remercier Mme Benbassa et ses collègues d'avoir suscité ce temps de débat. Bien que j'aie entendu votre annonce, monsieur le ministre, le Gouvernement ne me semble guère pressé d'inscrire à l'ordre du jour avec un temps de débat décent la proposition de loi dite « de lutte contre la maltraitance animale », issue de sa propre majorité.

Pour essayer d'éclairer notre débat de ce soir, je poserai deux questions. Premièrement, qui est opposé à un élevage respectueux des animaux associé à une rémunération équitable des éleveurs ? Deuxièmement, peut-on traiter une question aussi vaste et multidimensionnelle que l'élevage en deux heures d'examen

Il est maintenant convenu de parler de bien-être animal, expression consacrée administrativement et socialement. Il y a dans ce terme de communication une grande hypocrisie qui me gêne, mais c'est un autre débat. Essayons, avec modestie, de respecter les besoins fondamentaux des animaux que nous élevons pour les consommer ou consommer leurs produits ; ce sera déjà bien ! Quant à la seconde question,

que quelques-uns de ces éléments de complexité. Le premier est l'environnement européen, qui permettrait d'exporter dans notre périphérie ce qui serait interdit chez nous, par exemple le broyage des poussins et canetons ; c'est ce que j'appellerais l'exportation de la maltraitance. C'est donc une question européenne.

Enfin, j'ajouterai à ce très synthétique recensement de la complexité du problème la remise en question des grands accords de commerce international entre l'Europe et ses partenaires, de manière, là aussi, à éviter l'exportation de conditions d'élevage que nous n'accepterions plus chez nous.

construire un autre rapport à l'alimentation et aux animaux, qui soit éthique et représente un progrès moral de l'espèce humaine, tout en garantissant une alimentation saine et durable Cela suppose un énorme travail d'éducation, probablement sur plusieurs générations. En effet, ne nous leurrons pas : on ne change pas des comportements culturels aussi profondément ancrés que les comportements alimentaires en un claquement de doigts.

en imposant une surveillance vétérinaire, notamment par des outils vidéo, et par l'étourdissement préalable obligatoire, sans dérogation. Il est enfin en mesure de mettre en oeuvre les contrôles appropriés, notamment pour le transport et l'abattage.

L'alimentation, qui fut avec la protection contre les prédateurs la priorité de notre espèce, n'est plus que l'un des aspects de la consommation de masse. Il est temps de lui redonner toute son importance et, pour sa dimension animale, de l'inscrire dans le très nécessaire progrès moral de l'humanité. La discussion La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Il faut plutôt que le Gouvernement se mobilise sur le sujet, afin d'établir ce panorama précis et d'en faire une grande communication. Il est inutile d'inscrire ce genre de mesures dans la loi, puisque le Gouvernement peut déjà le faire. Notre avis défavorable

Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a demandé au Centre national de référence pour le bien-être animal de dresser un état des lieux des pratiques douloureuses en élevage, en vue de travailler sur des solutions Par ailleurs, la loi Égalim comporte plusieurs mesures visant à lutter contre la maltraitance animale, comme l'extension du délit de maltraitance animale aux établissements d'abattage et de transport d'animaux vivants, ou encore le doublement des peines.

pour l'avoir étudié dans votre rapport sur la détresse des agriculteurs. L'amendement a pour objet que, concrètement, la MSA active un accompagnement automatique en cas de confiscation du cheptel d'un agriculteur, événement traumatisant. Cette idée mérite d'être étudiée par le Gouvernement, comme le rapport le préconisait déjà, notamment son plan d'action et la convention d'objectifs et de gestion avec la MSA. Cela peut être mis en oeuvre dès demain,

Le Gouvernement partage la nécessité de sensibiliser les corps de contrôle à ces risques, en leur permettant, lorsqu'ils décident et exécutent une telle décision de confiscation, de délivrer une information complète aux agriculteurs concernés sur les aides psychologiques et économiques dont ils peuvent bénéficier. Le plan d'action devrait ainsi prévoir l'identification de référents départementaux économiques et sociaux, permettant de mieux coordonner les actions sur les territoires.

Pour ces raisons, et parce qu'il est pleinement mobilisé à travers ce plan d'action pour mener des actions spécifiquement en faveur des agriculteurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Comme l'explicite l'exposé des motifs, il s'agit d'un amendement d'appel, qui établit un lien très juste entre bien-être animal, bien-être des éleveurs

la prévention du mal-être et du risque suicidaire est un enjeu majeur des politiques publiques de santé au travail. S'appuyant, d'une part, sur le rapport du député Olivier sur les 63 recommandations formulées par la commission des affaires économiques du Sénat, dont les rapports étaient les sénateurs Ferrat et Cabanel, un plan d'action portant sur les moyens mis en oeuvre par l'État en matière de prévention et d'accompagnement des agriculteurs en situation de détresse sera présenté par le ministère de l'agriculture dans les prochaines semaines. Le plan de modernisation des abattoirs constitue également une formidable chance pour que les projets d'investissements améliorent réellement les conditions de travail

4. Mes chers collègues, je vous rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi,

Le groupe Les Républicains suivra l'avis de Mme la rapporteure, et cela pour plusieurs raisons. Les éleveurs français sont les premiers à être soucieux du bien-être de leurs animaux, et les méfaits de certains ne doivent pas jeter l'opprobre sur toute une profession.

intègre des critères de bien-être animal minimum- lumière, matériaux manipulables, abreuvement, etc. Ces évolutions sont également accompagnées par les consommateurs. C'est particulièrement visible pour les oeufs une baisse significative des capacités de production des élevages en cage a été constatée au profit des autres types d'élevages, lesquels représentent désormais 53 % des poules pondeuses, contre 19 % en 2008. Toutes ces avancées se sont faites sans recourir à la loi. Néanmoins, comme l'a expliqué Mme la rapporteure, la meilleure échelle pour prendre des décisions destinées à encadrer certaines pratiques d'élevage, de transport et d'abattage, comme le propose le texte,

favorable à l'adoption de ces quatre articles. Ce texte

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.